La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mardi 25 septembre 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté En application de l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2018-2019 est ouverte depuis le 1 octobre. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer des textes sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi et de la proposition de loi organique relatives à la lutte contre la manipulation de l'information ne sont pas parvenues à l'adoption de textes communs. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.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

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le pastoralisme est en danger. Croulant sous une avalanche de contraintes et exposé à une concurrence déloyale venue d'autres pays, l'élevage français pris globalement est en crise. Les éleveurs pastoraux ne sont pas épargnés par ces temps difficiles. Comme si leur métier n'était pas assez exigeant, leurs conditions de travail sont rendues toujours plus délicates par une succession de décisions défavorables, au premier rang desquelles celles qui favorisent la recrudescence des actes de prédation ! Les éleveurs pastoraux en ressentent dès lors un légitime sentiment d'abandon. Je crois que le Sénat entend leur détresse. C'est la raison pour laquelle il veut leur envoyer un signal fort. Un signal fort dont témoigne l'inscription de ce débat sur le pastoralisme en ouverture des débats de la session ordinaire. Un signal rendu encore plus fort par le fait que la proposition de résolution que nous examinons, déposée par Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, a été cosignée par plus de cent sénateurs venant de la quasi-totalité des groupes politiques, représentant tous les territoires. Cette prise de position sénatoriale transpartisane s'inscrit dans la continuité de travaux déjà engagés sur nos travées, tant au sein du groupe d'études Montagne, présidé par Cyril Pellevat, et du groupe d'études Chasse, présidé par Jean-Noël Cardoux, que du groupe de travail sur le pastoralisme dont j'assure la présidence et qui est rattaché à la commission des affaires économiques. Ces travaux ont vocation à se poursuivre, c'est essentiel pour nos éleveurs. La proposition de résolution qui nous est soumise est donc un coup d'envoi et non pas un coup de sifflet final.

les qualités sont trop souvent tues, est la vitrine de l'agriculture de demain. Dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier, une vingtaine de brebis ont été tuées dans le massif du Dévoluy. Jean-Claude Michel, président du groupe pastoral, est à bout, il n'en peut plus, la pression est vraiment trop forte, et surtout en ce mois de septembre Imaginez : 239 attaques dans les Hautes-Alpes depuis le début de l'année ! En ce 275 jour de l'année, je vous laisse faire le calcul : 36 jours sans attaque, alors que mon département a connu un hiver particulièrement rigoureux. C'est pour rappeler cette vérité qu'il était nécessaire que le Sénat prenne officiellement position sur le pastoralisme en rappelant toute l'importance qu'il a pour nos territoires. Car le pastoralisme est d'abord une question géographique. La question pastorale concerne très majoritairement les territoires montagneux, tant les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura que les massifs corses. Elle se pose aussi pour des littoraux du Nord, dans la baie d'Authie, pour les côtes normandes du Cotentin ou le delta camarguais au Sud. Elle concerne aussi l'estuaire de la Loire, les marais poitevins, ainsi que les prairies inondables de la Loire et de l'Adour. Elle s'invite même en zone périurbaine ! Presque tous les territoires sont concernés et le pastoralisme joue, du reste, un rôle primordial dans l'aménagement de nos territoires. Il suffit de songer à la contribution des producteurs à l'activité touristique, par exemple, grâce à la conservation des pistes de ski en montagne. Le pastoralisme exerce également un rôle en matière de prévention des risques naturels. En montagne, il permet de restreindre les risques d'avalanche, d'incendie ou de glissement de terrain. Le pastoralisme est aussi une question économique. C'est une pratique d'élevage qui concerne 14 000 fermes en France et près de 5 % du cheptel français. Dans les massifs montagneux, les pâturages collectifs utilisent parfois plus de 50 C'est une réalité que les politiques publiques doivent mieux appréhender, car les conditions d'exercice de ces métiers sont très particulières. C'est aussi une question agricole. Aux carrefours de toutes les attentes citoyennes, le pastoralisme promeut une agriculture extensive de qualité, à forte composante artisanale, souvent valorisée par le recours à des signes officiels de qualité. La question pastorale, c'est aussi une réponse aux défis environnementaux que nous avons à régler. L'élevage pastoral contribue au maintien des conditions essentielles à la préservation de la biodiversité, à la valorisation des ressources naturelles de nos territoires et à leur aménagement durable. C'est aussi une forme d'élevage qui prend en compte le bien-être animal puisque le cheptel est en semi-liberté et qu'il passe plusieurs jours dans les alpages durant l'estive, comme dans les Alpes. C'est enfin une question culturelle, puisque le pastoralisme s'exerce en France depuis des siècles et appartient au patrimoine français. Les images des grandes transhumances sont profondément ancrées dans l'esprit de nos concitoyens et sont, le plus souvent, au coeur de l'animation de la vie de nos régions rurales. Au fond, il s'agit de montrer que ces pratiques ancestrales sont très souvent modernes. En témoigne d'ailleurs l'attractivité du pastoralisme sur les jeunes agriculteurs. La résolution a pour objectif de rappeler tous ces éléments essentiels et de montrer aux producteurs concernés que les parlementaires considèrent la question pastorale dans son ensemble. Le pastoralisme ne se résume pas à la seule problématique de la prédation. Le champ est bien plus large. Au contraire, l'enjeu du débat est d'élargir l'horizon, de rappeler combien le pastoralisme est bénéfique à nos territoires, à l'environnement, à notre économie pour que le travail des éleveurs concernés soit reconnu à sa juste valeur. Toutefois, les auteurs de la proposition de résolution regrettent que les politiques publiques ne prennent pas en compte toutes ces spécificités de la question pastorale et toutes les externalités positives que le pastoralisme apporte à nos territoires et à notre économie. Ces effets positifs ne sont pas évalués à leur juste valeur. Un seul fait le démontre : les agriculteurs pastoraux ont un revenu trop faible au regard des conditions particulièrement difficiles de leur métier. À cet égard, il faut vivement regretter que les négociations relatives à la politique agricole commune, la PAC, puissent menacer encore leurs revenus à l'avenir. Ils sont également confrontés à des problématiques foncières et au renchérissement du prix des terres tendant à réduire les surfaces agricoles pastorales. La forêt s'étend, participant à ce rognage toujours plus inquiétant des surfaces pastorales. Dans ces conditions, et la résolution le rappelle, les éleveurs pastoraux se sentent laissés pour compte. C'est dans ce contexte déjà difficile que vient s'ajouter la problématique de la prédation. Pour les agriculteurs, la prédation a différentes formes- ours, loup, lynx -, mais elle concerne de plus en plus de territoires, compte tenu de l'expansion des zones de présence des loups. La détresse des éleveurs face à la multiplication des actes de prédation est immense et leur solitude dans ces épreuves, qui sont autant des drames économiques pour l'équilibre des exploitations que des drames humains, est profonde. Toutefois, les mesures déployées par l'État, notamment par le plan national d'actions Loup, ne sont pas à la hauteur de cette détresse. Quant aux élus locaux, ils sont confrontés aux conflits d'usage avec, par exemple, la problématique des chiens de protection qui attaquent les promeneurs, notamment dans les zones touristiques, le long des chemins de grande randonnée. Forte de cette série de considérations, la résolution émet deux séries de propositions. D'une part, elle appelle à valoriser à leur juste valeur les externalités positives induites par le pastoralisme. C'est une position conforme, je le crois, à une conviction profonde du Sénat, qu'il a exprimée à d'autres moments de manière unanime. Ce serait une grande avancée structurelle pour les agriculteurs concernés. invite également, à plus court terme, à sanctuariser les moyens accordés à l'agriculture pastorale, notamment dans les négociations en cours sur la PAC. Les éleveurs pastoraux ne sauraient être les grands oubliés du second pilier D'autre part, la résolution demande la rénovation urgente de la politique relative au retour des grands prédateurs sur nos territoires. Sur la problématique de l'ours, elle appelle à ce que toute réintroduction d'ours ne se décide pas unilatéralement dans un bureau parisien, mais soit bien précédée d'une étude d'impact exhaustive et d'une concertation préalable avec les éleveurs et les élus locaux. les loups, elle appelle à suivre trois axes de travail, reprenant en cela les travaux du groupe d'études Montagne sur le loup réalisés il y a quelques mois. Premièrement, il faut améliorer la connaissance de la situation actuelle en fiabilisant les données sur le nombre de loups à destination des élus locaux et en renforçant les connaissances scientifiques sur l'hybridation et le comportement des loups. Deuxièmement, il convient de réapprendre aux loups à se tenir à l'écart des hommes et des troupeaux par le recours à des méthodes alternatives complémentaires aux tirs de prélèvement. Troisièmement, la résolution précise que le système d'indemnisation des éleveurs est insuffisant aujourd'hui. Les paiements doivent être accélérés et mieux prendre en charge les chiens de protection. Le choix du Gouvernement de conditionner les indemnisations à la mise en place de mesures de protection doit être questionné, tout comme doivent être mieux reconnus les troupeaux non protégeables. Pour conclure, il me semble que cette résolution permet d'envoyer un message fort à tous les agriculteurs pastoraux français. Elle témoigne du soutien qu'ils trouveront toujours chez les parlementaires représentant les territoires. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, est une espèce « strictement protégée », inscrite à l'annexe II de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée en 1979 et ratifiée par la France en 1990, mais aussi aux annexes II et IV de la directive européenne de 1992 dite « Habitats-faune-flore », où il est classé « prioritaire d'intérêt communautaire Cette politique a entraîné une réintroduction du loup sur le continent européen. Depuis le milieu des années 2000, la filière de l'élevage est confrontée à une forte augmentation des attaques de loups sur les troupeaux. En dix ans, le nombre de bêtes tuées en France est passé de 2 500 en 2007 à 12 12 000 en 2017. Le nombre d'exploitations ovines est, en revanche, passé de 95 000 en 2010 à 70 000 en 2016. Les éleveurs d'ovins saisissent de plus en plus fréquemment les élus et les services de l'État de la multiplication des attaques et des prédations. Selon les professionnels, le préjudice s'élèverait à 26 millions d'euros. Si le nombre de meutes de loups est difficile à estimer, il paraît avoir augmenté de manière significative compte tenu des témoignages et de l'accroissement du nombre d'attaques. De même, le comportement du loup envers les humains est potentiellement modifié par son hybridation avec des chiens, fait insuffisamment pris en compte à l'heure actuelle. Cet accroissement des attaques de troupeaux ne paraît pas maîtrisé et menace l'activité des bergers et éleveurs qui entretiennent avec passion des centaines de milliers d'hectares de biodiversité. Dans les zones de montagne, les éleveurs participent à la richesse écologique et économique des territoires. Le pastoralisme et Le pastoralisme et l'élevage extensif sont des piliers de la biodiversité et de la vie rurale qui sont les derniers remparts contre la déprise, l'embroussaillement et les incendies ravageurs. le plateau du Larzac- et un petit peu dans les départements de la Lozère, du Gard et de l'Hérault -, l'agropastoralisme s'est beaucoup développé, permettant d'assurer une biodiversité remarquable, qui justifie que cette petite région soit classée à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des milliers de brebis y entretiennent des centaines de milliers d'hectares de biodiversité. La présence du loup et les attaques répétées découragent nos éleveurs de sortir avec les animaux. Ainsi, si rien n'est fait, si aucune solution n'est trouvée, nos paysages vont s'embroussailler et mettre fin à cette biodiversité qui voit actuellement de nombreux touristes d'Europe du Nord venir, aux mois de mai et juin, photographier nos orchidées et nos plantes rares. Aujourd'hui, les éleveurs demandent la révision de la convention de Berne pour deux raisons. D'une part, le loup n'est, au vu des chiffres, plus menacé en Europe : on en compterait 20 000 sur le continent. D'autre part, il semble que les loups « hybrides » soient à l'origine de la plupart des attaques de troupeaux. Or la convention de Berne ne distingue pas les « vrais » loups des « hybrides

Nous ne pouvons plus l'ignorer, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Pologne ou en Roumanie ! La position de l'Union européenne consiste à considérer que la cohabitation entre loups et élevages fonctionne convenablement, que les outils techniques comme les portails électriques sont efficaces. Il ne resterait qu'à convaincre des éleveurs

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la cohabitation « heureuse »- puisque c'est un terme qu'on emploie souvent ! -avec le loup n'existe pas, c'est un mythe ! Elle provoque le désarroi et se fait au prix d'un fort recul de l'élevage et d'une diminution de la biodiversité. La réglementation européenne relative au statut de protection des loups doit évoluer pour que le pastoralisme que nous défendons ne disparaisse pas au profit de l'élevage industriel hors-sol qui, lui, n'a rien à craindre des loups Les prélèvements de loups doivent s'effectuer en fonction des dégâts aux troupeaux et non dans un cadre de gestion de l'espèce contraint par la directive Habitats et la convention de Berne. En outre, on peut s'interroger sur l'efficacité et la capacité réelle de la brigade loup ! Comment une seule brigade d'intervention de douze personnes basée dans le Sud-Est peut-elle couvrir les presque vingt-cinq départements concernés ?

chers collègues, l'actualité ne cesse de nous rappeler la vulnérabilité du monde pastoral. Il y a quelques jours, la brigade loup a d'ailleurs été dépêchée dans les Pyrénées-Atlantiques, en vallée d'Ossau, pour protéger les éleveurs face à la prédation du loup. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et le groupe d'études Développement économique de la montagne, que j'ai l'honneur de présider, sont particulièrement attachés à la défense du pastoralisme et des éleveurs. Face aux inquiétudes suscitées par le plan Loup présenté par le Gouvernement le 19 février dernier, la commission m'a confié, et j'en remercie son président Hervé Maurey, la mission d'établir rapidement un diagnostic et des préconisations pour répondre au malaise grandissant du monde pastoral. Le rapport adopté en avril par notre commission formule ainsi quinze propositions, reprises très largement dans la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui. Ces propositions ne constituent pas une remise en cause de la présence du loup dans notre pays. J'insiste : il s'agit avant tout d'apporter une vision apaisée sur ce sujet, où les passions s'expriment parfois de façon vigoureuse et pas suffisamment rationnelle. Aussi ce rapport invite-t-il l'ensemble des services concernés de l'État à renforcer la fiabilité et la fluidité de l'information concernant le nombre de loups, à mieux protéger et accompagner les éleveurs face à la prédation et à revoir globalement la gestion des loups, en améliorant la connaissance de leurs comportements et les mesures alternatives aux tirs de prélèvement, par exemple. Dans le prolongement de ces travaux, je souhaiterais saluer l'initiative de notre collègue Patricia Morhet-Richaud, qui a souhaité nous associer, Jean-Noël Cardoux et moi-même, à l'écriture de cette proposition de résolution sur le pastoralisme, déposée par la présidente Sophie Primas, à la suite du voeu que le président Gérard Larcher a exprimé. Au-delà, je souhaite vous remercier, mes chers collègues, d'avoir très largement répondu à l'appel en cosignant cette proposition de résolution ou en lui apportant votre soutien. Cette initiative prolonge d'ailleurs la mobilisation de nombre de nos collègues, alertés depuis longtemps par les élus, les éleveurs et la population et je et je me réjouis du caractère transpartisan de nos travaux sur le sujet. S'agissant du texte de la proposition de résolution dont nous avons à connaître, je souhaiterais insister sur deux points. D'abord, Patricia Morhet-Richaud l'a rappelé, si le pastoralisme contribue largement au maintien de la biodiversité dans notre pays, il est exposé à des dangers mortels, près de cinquante ans après l'adoption de la loi pastorale de 1972. Alors que nous parlons de transition écologique, de biodiversité, de meilleurs usages alimentaires, nous sommes précisément en présence d'une activité qui répond à ces objectifs. Les éleveurs sont davantage que des gardiens des montagnes et des plaines, ce sont les premiers écologistes Ils ne consomment pas- ou peu - de produits chimiques et l'élevage extensif assure à la fois la protection du sol, de l'eau et contribue à l'entretien des paysages. Il figure, à ce titre, parmi les bonnes pratiques pour la gestion des sites Natura 2000. Aussi, au regard de la relative passivité des pouvoirs publics face à la disparition progressive des oiseaux ou d'autres espèces animales comme les abeilles, leur attitude concernant les prédateurs et le pastoralisme apparaît-elle excessive et déséquilibrée. Ensuite, il est aujourd'hui clair que l'équilibre entre la protection des prédateurs- en particulier celle du loup au titre de la convention de Berne et du code de l'environnement -et le maintien de l'agropastoralisme est défavorable aux éleveurs. Les chiffres sont éloquents : 11 000 victimes animales du loup en 2017, en augmentation de 60 % depuis 2013 et une dépense publique consacrée à la prédation du loup qui est passée de 4 millions d'euros en 2006 à 26 millions d'euros en 2017, sans compter les moyens humains et le temps consacrés à la gestion des dégâts causés par le loup Nous assistons donc à la faillite du modèle de cohabitation entre le loup et l'élevage tel qu'il est pensé depuis vingt ans en France. Qui plus est, nous sommes en train de perdre la bataille de la communication face à une pensée urbaine de la ruralité qui empêche d'apporter des solutions concrètes et pragmatiques. Monsieur le ministre, pour avoir rencontré à de nombreuses reprises des membres de votre cabinet, je sais que vous êtes attentif à ce sujet et nous serons à vos côtés, comme à ceux des éleveurs. Aussi, je vous invite, mes chers collègues, à voter cette proposition de résolution pour envoyer un message clair à l'ensemble des acteurs directement concernés par l'avenir du pastoralisme. Les éleveurs et les territoires pastoraux ne peuvent attendre davantage ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'économie pastorale constitue un élément incontournable du modèle agricole français. Le modèle d'élevage extensif appartient à notre patrimoine et il est de notre devoir, en tant que sénateurs et représentants des territoires, de nous mobiliser afin de sauvegarder cette tradition culturelle ancestrale. Nous le savons, les gains résultant pour les milieux naturels de la pratique du pastoralisme sont considérables et bénéficient à toute la société. Je citerai, à titre d'exemple, l'aménagement des territoires et le façonnement de nos paysages profitant particulièrement au secteur du tourisme, ainsi que la protection de la biodiversité- le pastoralisme constitue depuis toujours un véritable mode de gestion restauratoire utilisé pour l'entretien et la restauration des milieux naturels. Enfin, l'agriculture pastorale, caractérisée par une forte composante artisanale, favorise la production de denrées alimentaires de qualité, souvent valorisées par le recours à des signes officiels de qualité et aux circuits courts. Depuis une vingtaine d'années, nous observons une augmentation substantielle du nombre de loups qui colonisent les espaces pastoraux, engendrant une préoccupation légitime de la part du monde pastoral. Il est certain qu'une refonte du modèle de gestion du loup est nécessaire pour accompagner et moderniser le pastoralisme. Elle offrira aux éleveurs des perspectives d'avenir crédibles pour leurs métiers, pour leurs produits et pour leurs partenaires territoriaux. C'est ce à quoi s'est attaché le Gouvernement par l'établissement du plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage. Mes chers collègues, deux objectifs doivent nous animer tout au long de ce débat et, je le crois, ils ne sont en rien incompatibles d'une part, le maintien de nos écosystèmes par la protection des différentes espèces de prédateurs ; d'autre part, la pérennisation du modèle agricole pastoral. La préservation de la biodiversité dans nos territoires ne doit certainement pas négliger la contribution du pastoralisme au maintien des écosystèmes floristique et faunistique, elle ne peut se faire au détriment du soutien au retour de certains grands prédateurs. Venons-en à la proposition de résolution : je tiens à saluer le travail effectué en amont de ce texte par notre collègue Cyril Pellevat l'année dernière. Toutefois, par cette proposition de résolution, mes chers collègues, vous tendez à opposer la refonte du dispositif de gestion du loup à la défense des intérêts des éleveurs du monde pastoral. Pourtant, il me semble que l'action du Gouvernement propose des solutions visant à assurer la viabilité de l'espèce en France tout en protégeant mieux les troupeaux et les éleveurs. Le plan ne constitue pas, comme j'ai pu le lire, une succession de mesures antipastorales. C'est incroyable ! Il est le fruit d'une consultation riche en enseignements et élabore une nouvelle méthode de gestion du loup fondée,

De nouvelles mesures significatives sont mises en oeuvre pour la protection des troupeaux face aux attaques et pour mieux aider les éleveurs à se défendre.

un encadrement plus efficace des modalités de gestion des tirs d'effarouchement, de défense et de prélèvement. le plan prévoit de soutenir l'élevage et le pastoralisme dans les zones de présence du loup par une meilleure aide à l'emploi, un soutien important aux filières de produits agricoles de qualité et par de réelles mesures d'amélioration des conditions de vie des bergers. Ce plan national d'actions adopte le principe d'une gestion adaptée aux impacts sur l'élevage et aux réalités du territoire. Les effets des mesures mises en oeuvre seront pris en compte afin de réaliser des actions pertinentes sur le terrain. Par ailleurs, certains d'entre vous ont manifesté leur inquiétude concernant la tournure des négociations en cours de la politique agricole commune. Mes chers collègues, faisons confiance au ministre de l'agriculture pour défendre les intérêts de nos éleveurs Au regard des solutions apportées par le plan Loup de l'année dernière, dont l'évaluation à mi-parcours conditionnera la mise en place de la deuxième phase,

Ce mode d'élevage respectueux des animaux prévient des risques naturels, protège les écosystèmes et accompagne les autres activités humaines. Il est tout simplement indispensable à la vie de nos montagnes, et nous devons tout faire pour le préserver. Malheureusement, sa situation se dégrade de manière structurelle, et cela pour plusieurs raisons : la rudesse du métier, une crise des vocations, les difficultés économiques du monde agricole et, comme cela a été rappelé, la concurrence déloyale à travers les traités de libre-échange, la raréfaction du foncier, une forte dépendance aux fragiles subventions européennes, le réchauffement climatique et la sécheresse. Le retour des grands prédateurs, particulièrement du loup, est venu noircir ce tableau déjà alarmant. La détresse et le sentiment d'impuissance des éleveurs grandissent, et il nous faut y répondre impérativement. Mais, comme tentent de le faire cette proposition de résolution et le plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage, c'est de manière globale qu'il faut appréhender le problème. Aussi, nous partageons les constats, les considérants et la plupart des invitations au Gouvernement que formule cette proposition de résolution, en particulier la nécessité de sanctuariser les zones de pâturage de type garrigue ou maquis dans le périmètre des aides la nécessité d'améliorer la connaissance scientifique de l'éthologie du loup pour proposer des modes de protection des troupeaux mieux adaptés. Monsieur le ministre, le plan Loup porte les germes d'une véritable politique pastorale que nous appelons de nos voeux. Le Gouvernement doit maintenant s'engager sur des moyens financiers suffisants pour développer les brigades loup, recruter des aides-bergers, accompagner le dressage des chiens de protection, indemniser promptement et justement les éleveurs, les accompagner après le traumatisme d'une attaque et conduire les recherches nécessaires sur le prédateur. À ce jour, les moyens annoncés nous semblent insuffisants. Je m'inscris d'ailleurs en faux contre le discours trop souvent entendu- notamment sur les travées de la majorité sénatoriale -bien qu'il soit absent de ce texte, selon lequel le loup coûterait trop cher. C'est trop vite oublier qu'entre la moitié et les trois quarts des 26 millions d'euros du plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage sont directement attribués aux activités d'élevage comme l'embauche, notamment d'aides-bergers. On ne peut pas, dans le même temps, dénoncer des moyens insuffisants et reprocher à l'État de trop dépenser. À titre de comparaison, on rappellera que les seules indemnisations des agriculteurs victimes des sangliers s'élèvent à environ 50 millions d'euros par an. L'heure est pourtant grave et appelle une mobilisation générale pour la préservation du pastoralisme et de la biodiversité. Pour cette raison, nous voterons en faveur de cette proposition de résolution que nous avons pu amender quelque peu. Nous émettons toutefois une réserve importante. Si une réflexion à l'échelle européenne est indispensable, l'invitation à réviser le niveau de protection des grands prédateurs à l'échelle européenne et internationale n'est pas acceptable et ne peut représenter une solution viable. Entendons-nous bien : nous comprenons tout à fait la nécessité d'abattre un animal pour protéger un troupeau et prenons la pleine mesure de la nécessaire régulation à mettre en place, mais ce n'est pas faire justice au pastoralisme que de considérer, comme le font certains, que son salut passera par l'extermination des prédateurs. C'est un miroir aux alouettes, un message facile que l'on propose aux éleveurs. Un tel combat international mobiliserait une énergie et un temps considérables sans aucune garantie de réussite. C'est autant de temps et d'énergie qu'on ne consacrera pas à travailler à l'inévitable et nécessaire cohabitation entre prédateurs et troupeaux. Même dans le cas, improbable, où la chose serait autorisée, exterminer les prédateurs sur notre sol ne serait pas une mince affaire. Durant des siècles, nous avons tenté de chasser le loup. Nous avons pour ce faire mobilisé des milliers d'hommes- y compris l'armée sous l'Empire -, et nous avons brûlé des milliers d'hectares de forêt.

De la même manière, nous le savons, il n'est pas beaucoup plus simple de contenir la surpopulation de sangliers, espèce pourtant non protégée qui ravage nos cultures. Comme nos voisins européens, accompagnons la cohabitation. L'enjeu consiste à la fois à mieux protéger les troupeaux et à mieux accompagner les éleveurs avant et après les attaques. Il est également indispensable de développer des modes de protection alternatifs et de tester de nouvelles techniques d'effarouchement, telles que les tirs non létaux ou le piégeage. Dans les territoires en recherche de réponses concrètes des initiatives se mettent en place. Je pense, par exemple, au projet d'expérimentation du parc naturel régional du Vercors, que je vous invite d'ailleurs à soutenir, monsieur le ministre. Après plusieurs mois de concertation avec tous les acteurs concernés, éleveurs, associations environnementales, élus, services de l'État, le parc a adopté à l'unanimité, le 19 septembre dernier, un plan d'action visant à mieux protéger les troupeaux, à soutenir l'activité pastorale et touristique et à permettre une cohabitation la plus raisonnable possible avec le loup. C'est le projet le plus équilibré, le plus efficace et le plus honnête à proposer à nos éleveurs. C'est le moyen le plus sûr pour sortir des postures en agissant sans attendre pour préserver le pastoralisme. Cette résolution formulant de nombreuses propositions dans ce sens, nous la voterons en dépit de nos réserves. Il est important de sortir de l'affrontement stérile sur le loup ou l'ours et de parler d'une seule voix pour défendre le pastoralisme et la biodiversité. Très

s'ouvrent sur le thème du pastoralisme, donnant ainsi la parole aux territoires ruraux et de montagne. Notre Haute Assemblée assure ainsi pleinement la mission de représentation des territoires de la République que lui confère la Constitution. Département rural s'il en est, mon département de l'Ariège est aussi un département pastoral. L'estive qui est pratiquée dans plus de 50 % des exploitations n'a pas seulement une vocation productiviste, loin de là, mais remplit surtout une mission d'entretien de la montagne par les troupeaux. Le pastoralisme ariégeois qui s'étend sur 115 000 hectares, soit 25 % du territoire du département, a pour spécificité principale de s'exercer sur des terres ouvertes à tous. cette activité s'exerce à 90 % sur des espaces qui appartiennent soit à l'État, soit aux communes. C'est en quelque sorte l'essence même du pastoralisme, qui se matérialise par des modes d'appropriation et de gestion collectifs au sein d'espaces semi-naturels spécifiques extensifs, où règne une biodiversité incomparable. À l'heure où la mode est au « produire local », où les Français sont prêts à consentir un effort financier parfois important pour certains foyers afin de se nourrir avec une alimentation de qualité issue de circuits courts, une production « de la fourche à la fourchette », notre devoir est d'encourager le développement de ces modes de production totalement naturels pour lesquels la traçabilité est garantie au consommateur. Après avoir connu une démographie en baisse durant près d'un siècle, la courbe aurait tendance à s'inverser et nos territoires, entretenus par l'activité de l'homme, qu'elle soit à vocation pastorale, agricole, forestière ou touristique, redeviennent des milieux ouverts et accessibles. Nous le savons, sans cette présence humaine, ce sont des sentiers qui se ferment, des paysages qui s'ensauvagent alors qu'ils sont si riches quand ils sont sillonnés par les troupeaux. Aujourd'hui les bergers pyrénéens sont exaspérés et abattus, car ils sont confrontés à une augmentation sans précédent des dommages causés par des prédateurs, et plus précisément par les ours.

Au 31 août de cette année, on dénombrait 232 attaques, soit 30 % de plus par rapport à l'année précédente, et déjà 372 victimes, alors que tous les troupeaux ne sont pas encore redescendus dans les vallées. Pourtant une nouvelle réintroduction d'ours slovènes est annoncée pour les semaines à venir sans qu'aucune concertation ait été organisée. Un travail commun et préalable avec l'État est fondamental, monsieur le ministre,

les autorités doivent « assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l'ours dans les territoires exposés à ce risque ». Nous le savons, les mesures de protection traditionnelles avec les chiens de protection ou la création de parcs de nuit ne suffisent plus, car l'ours a appris à les déjouer. Il faut trouver d'autres mesures d'accompagnement afin de mieux protéger les biens des éleveurs, leurs troupeaux, mais aussi les maires qui pourraient voir leur responsabilité pénale engagée en cas d'attaque mortelle dans leur commune.

Si nous ne réagissons pas, nous prenons le risque de voir une profession entièrement découragée et de mettre à mal, non pas l'agriculture industrielle, mais l'agriculture de qualité, cette agriculture paysanne qui se nourrit du pastoralisme dont j'ai essayé de rappeler tous les précieux services économiques, environnementaux et culturels qu'il nous rend. Cessons d'avoir une approche romantique de l'ours pour nous tourner vers une approche pragmatique ! Nos montagnes doivent rester le théâtre d'une biodiversité que nous appelons tous de nos voeux, des montagnes vivantes, avec des hommes et des femmes qui y habitent et y travaillent au quotidien, des montagnes également profitables à ceux qui y séjournent quelques jours par an et qui m'ont inondé de SMS avant que je ne monte à cette tribune. Pour toutes ces raisons, mon groupe soutient dans sa grande majorité cette proposition de résolution sur le pastoralisme

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier M. le président du Sénat ainsi que les membres du groupe de travail sur le pastoralisme et notre collègue Patricia Morhet-Richaud d'avoir aujourd'hui voulu mettre en lumière le pastoralisme, aborde la problématique de cette pratique ancestrale avec réalisme, respect des hommes, des cultures et des modes de vie. Elle met l'accent sur les difficultés des éleveurs aux pratiques vertueuses qui, au-delà d'une économie favorisant l'excellence, protègent une vie touristique, garantissent le maintien des populations montagnardes, la lutte contre la fermeture des milieux et la préservation d'un environnement souvent soumis à des aléas climatiques violents. Monsieur le ministre, je sais que vous connaissez bien le département des Hautes-Pyrénées. Lors de leur congrès en juin dernier, les jeunes agriculteurs vous ont expliqué les difficultés et les particularités de la pratique du pastoralisme. Vous avez entendu leur cri d'alarme. Alors que nous travaillions sur cette proposition de résolution, l'actualité nous a rattrapés avec l'annonce, par le ministre de la transition écologique et solidaire, de la réintroduction de deux ours en Béarn et de la réactivation du plan Ours. Comment comprendre une telle décision qui fragilise toute une profession déjà affaiblie ? Comment peut-on sacrifier toute une économie à un choix idéologique ? Quel sera l'avenir de nos montagnes ? Deviendront-elles un espace réservé aux prédateurs dont on aura chassé toute présence humaine ? Ce n'est pas notre choix. Comment peut-on imposer aujourd'hui à des éleveurs déjà harassés de travail de monter à plus de 2 000 mètres d'altitude tous les soirs pour garder leurs troupeaux ? Comment peut-on aujourd'hui leur rajouter des contraintes et de la peur ? Depuis les premières réintroductions d'ours dans les Pyrénées, force est de constater qu'aucune des mesures d'accompagnement mises en place n'a fonctionné. Il y a aujourd'hui une réelle incompatibilité entre la présence de grands prédateurs et celle des troupeaux. Va-t-on persister dans ces erreurs ? Va-t-on enfin écouter la voix unanime des parlementaires de ces territoires ? Allez-vous aujourd'hui entendre cette proposition de résolution de la Haute Assemblée qui se dresse pour préserver les territoires ? J'ai eu l'occasion de dire au ministre François de Rugy que, par ces mesures, il expose le pastoralisme à une mort certaine. Face à cette situation, nous ne pouvons nous résigner. Cette proposition de résolution est un cri d'alarme, une alerte de nombreux élus de montagne qui s'inquiètent face au désarroi de leurs éleveurs. Elle vise à replacer cette économie, son savoir-faire et ses bienfaits au centre de nos préoccupations. Monsieur le ministre, je sais que vous n'êtes pas responsable de ces réintroductions, mais vous avez le devoir de prendre en compte cette détresse et de défendre cette profession. Vous avez le devoir de prendre en considération les demandes légitimes d'études d'impact et de concertation avec les populations concernées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant qu'élue des Pyrénées-Atlantiques où la réintroduction de l'ours est plus que jamais un sujet de préoccupation pour nos éleveurs pastoraux, j'accueille avec enthousiasme cette proposition de résolution. Bien qu'elle n'ait pas d'effet contraignant, elle permet d'acter la prise en compte par le Sénat de la désespérance du monde pastoral et permettra, je l'espère, de donner de l'écho à son message.

prédateurs et le pastoralisme suscite des inquiétudes légitimes pour les acteurs économiques de nos montagnes. Il est vrai que les consultations menées donnent le sentiment que la concertation n'était qu'un déroulé en bonne et due forme et obligatoire de la procédure administrative, mais qu'au fond, la décision était déjà prise. Tout cela ne peut qu'engendrer de la défiance. Entre sentiment d'incompréhension et d'abandon, le monde pastoral vit cette période comme un ajout supplémentaire de difficultés à un métier déjà difficile et exposé à une avalanche de contraintes impacts du changement climatique, compétition internationale, crise des vocations, poids des normes, recrudescence des actes de prédation ... La liste est longue et incomplète.

de s'acheminer vers une agriculture plus qualitative que quantitative. Les éleveurs qui perpétuent cette tradition culturelle, élaborent des produits de haute qualité artisanaux et permettent des externalités positives n'ont-ils pas toute leur place dans cette vision de l'agriculture ? Je partage bien entendu tous les constats et les objectifs de cette proposition de résolution, mais je voudrais insister sur un point particulier. Il me semble qu'il faut aller encore plus loin que la refonte du système d'indemnisation des éleveurs, qui ne constitue qu'un seul des volets du traitement de cette problématique. Développer l'attractivité du métier d'éleveur me semble un moyen de redonner du sens et de la dimension. Nous ne voulons pas de territoire sanctuarisé, mais des territoires vivants dans lesquels l'homme a toute sa place. Pour cela l'économie de montagne doit être préservée et encouragée. L'État doit savoir accompagner de manière spécifique les territoires dans lesquels il a décidé de de réintroduire l'ours ou le loup. Je pense par exemple au suivi de ces grands prédateurs par GPS. L'État doit être performant et partager cette technologie avec les éleveurs afin de permettre la localisation de ces animaux et de prévenir les attaques des troupeaux. Les conditions de vie des éleveurs doivent également être repensées tout en tenant compte des aspirations et des exigences de notre temps. Cela peut se traduire par des moyens de transport, comme le quad, leur permettant de rejoindre plus facilement les estives depuis la vallée. En conclusion, mes chers collègues, au gré des réintroductions d'ours et de loups dans nos territoires, j'encourage le Gouvernement à préserver le pastoralisme et à apporter des réponses pragmatiques et respectueuses des hommes et des femmes qui vivent et qui travaillent dans les zones impactées. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui est un signal fort pour les territoires pastoraux et pour l'ensemble des éleveurs alors que la cohabitation entre le loup, l'homme et les activités d'élevage se dégrade considérablement. me l'a dit récemment, l'histoire du loup a changé son métier. Dans les Alpes-Maritimes où l'élevage ovin est réalisé en estive presque toute l'année, c'est la survie du pastoralisme qui est engagée, sachant que mon département détient le record du nombre d'attaques- près de 3 000 en 2016. Alors que les troupeaux comptaient jusqu'à 100 000 bêtes il y a vingt-cinq ans, l'effectif actuel est tombé à 30 000 avec, en parallèle, l'expansion continue du prédateur dans tout l'arc alpin depuis 1992. 1992. Mes collègues du groupe Les Républicains et moi-même pensons, comme les bergers, que le chiffre officiel de 430 loups sur le territoire national s'avère très en deçà de la réalité,

à ce qu'a dit notre collègue Guillaume Gontard, nous ne voulons pas l'éradication du loup, mais nous souhaitons arriver à une plus grande régulation de la population. Dans ce contexte, la déception vis-à-vis du plan Loup fut à la hauteur des espoirs suscités par les propos du Président de la République qui, un mois plus tôt, lors de ses voeux aux agriculteurs, avait annoncé vouloir « remettre l'éleveur au milieu de la montagne », de manière à ce que le plan Loup « soit fait et pensé dans les territoires où on le décline ». Cette volonté était partagée par l'ensemble des éleveurs, des organisations agricoles et des élus des départements concernés qui pensaient que le Gouvernement avait enfin compris que seules des décisions pragmatiques courageuses et ambitieuses répondraient aux attentes accumulées en vingt-huit ans. Mais, après cette occasion manquée, les éleveurs ont la sensation que leur voix ne compte pas

alors même que sont refusés des permis de construire pour des bergeries en dur et que les chiens patous sont eux aussi massacrés par les loups -et, d'autre part, d'un préjudice moral qui est loin d'être anecdotique. Les éleveurs les plus pessimistes pensent qu'il est déjà trop tard pour agir. Pourtant, un moyen simple serait de multiplier le nombre de brigades loup localement, afin d'en faire un véritable outil au service des collectivités qui relèvent les plus forts taux d'attaques. À ce sujet, les interrogations sur la pérennité de la brigade loup dans le temps et la possibilité pour les collectivités locales de prendre l'initiative d'en créer reste d'actualité. En effet, si vous m'aviez confirmé, monsieur le ministre, la pérennisation des emplois, le précédent ministre de la transition écologique et solidaire avait fait naître un doute en précisant : « Toutefois, cette formation qui représente un engagement financier conséquent, ne pourra être étendue à toutes les régions où le loup est implanté.

pour que perdurent les activités de pastoralisme, une réflexion devra aussi être menée sur la suspension temporaire du nombre de loups à abattre, car le fameux quota annuel de destruction de loups montre toutes ses limites. D'une part, l'estimation administrative en amont ne répond pas aux besoins- ce fut le cas en 2017, au point que Nicolas Hulot avait dû augmenter en urgence le quota d'abattage, compte tenu de la menace de prédation -et, d'autre part, la méthode des tirs isolés de prélèvement semble fixer une limite à ne pas dépasser sans répondre à un objectif de préservation du pastoralisme. Plutôt que de proposer de nouvelles mesures accessoires aux départements les plus touchés,

aux situations déjà identifiées dans les départements. Nous savons que les dommages pastoraux ne se répartissent pas de façon uniforme en France, mais reflètent deux phénomènes distincts d'un côté, des attaques graves, concentrées notamment dans les villages des Alpes-Maritimes, dont certains n'ont jamais connu de répit depuis 2002, et de l'autre, des attaques sporadiques dans des territoires plus vastes où la présence du loup est récente. Il faudra donc avoir le courage, pour assurer la survie des activités de pastoralisme,

dont 40 % dans les seules Alpes-Maritimes. Les éleveurs veulent simplement exercer leur métier en toute sécurité, mais face à un ensauvagement qui fait courir un risque sérieux au pastoralisme,

Depuis un siècle, la société a beaucoup évolué et le pastoralisme s'est considérablement transformé. Aujourd'hui ce système fait partie intégrante du développement rural et assure ainsi une multifonctionnalité qui n'est plus à remettre en cause. C'est une source d'emplois diversifiés, permanents ou saisonniers, qui renforce un ancrage territorial, vecteur de lien social. Ce système est reconnu pour favoriser des pratiques d'élevage qui permettent de maintenir des paysages ouverts et accueillants, favorables à la biodiversité. Le pastoralisme est reconnu également parmi les systèmes productifs les mieux-disants en termes de multiperformance écosystémique et de développement durable parmi toutes les autres productions agricoles. Face au changement global et irréversible du climat, et selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, « les pelouses d'attitude sont un des écosystèmes français stockant le plus de carbone les prairies permanentes gérées de manière extensive « présentent en général un bilan global beaucoup plus intéressant que les surfaces cultivées puisqu'elles constituent des puits nets en termes de captage de CO2 ». De même, la contribution du pastoralisme à la limitation du risque d'incendie et d'avalanche n'est plus à démontrer. L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, précédemment évoquée par l'un de mes collègues, des paysages culturels de l'agropastoralisme des Causses et des Cévennes démontre la valeur universelle du pastoralisme. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui souligne largement ces points forts, mais aussi les difficultés rencontrées par le pastoralisme et ses acteurs. L'un des enjeux forts auxquels nous devons répondre est celui du revenu de ces agriculteurs, structurellement inférieur à la moyenne de la profession. C'est pourquoi il est primordial de prendre en compte et de soutenir les dynamiques collectives- les mesures agroenvironnementales, ou MAE, et les systèmes herbagers pastoraux -avec un mécanisme de plafonnement adapté, en privilégiant par exemple l'emploi.

et, de l'autre, des agriculteurs peu soucieux de leur environnement. Les bergers sont aussi préoccupés par le bien-être de leurs animaux. Ils ne nous parlent pas que de rendement, mais aussi de moutons voués au grand air,

Caricaturer le débat ne peut en aucun cas permettre d'y apporter les bonnes réponses. Au contraire, il nous faut favoriser les temps de concertation, les diagnostics, les équipements qui permettront de concilier activité pastorale et autres activités. Les attentes sont grandes et les enjeux importants. Il est à espérer que cette proposition de résolution pourra servir de base à un renforcement de la politique nationale de soutien au pastoralisme et à sa meilleure prise en compte dans le cadre de la future PAC. je m'associe aux propos de mon collègue Alain Duran concernant la position de mon groupe pour le vote de cette proposition de résolution. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviens en tant que signataire de la proposition de résolution sur le pastoralisme.

national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage repose sur un principe d'équilibre entre la conservation des espèces et la prise en compte de la détresse des éleveurs. Or cet équilibre n'existe pas,

Il faut souligner que seuls les animaux mordus figurent parmi les victimes, alors que des moutons meurent en sautant des barres rocheuses pour échapper aux canidés et que nombre de brebis avortent, stressées par les attaques, ce qui augmente le nombre réel de victimes. De même, cette coexistence n'est plus pacifique parce que les loups eux-mêmes ont changé. Un travail d'enquête publié dans mon département, en janvier 2017, par l'INRA et le Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée démontrait déjà que les loups franchissaient la lisière des forêts et se rapprochaient de plus en plus des habitations humaines. Ces animaux « s'adaptent, évoluent en fonction de nous », expliquait le chercheur Michel Meuret. Mes chers collègues, la vocation des bergers n'est ni de tuer des loups ni de se transformer en éleveurs professionnels de chiens d'Anatolie ou de patous, non plus que de monter des dossiers pour solliciter des subventions destinées à compenser la perte de leurs bêtes. Que des bergers désertent certains espaces parce qu'il est impossible de préserver leur troupeau, voilà une très mauvaise nouvelle pour l'environnement montagnard, qu'ils ne pourront plus entretenir.

faute de bergers présents ? Voulons-nous pleurer des zones entières carbonisées, comme en Californie ? Enfin, il faut aussi prendre en compte le désarroi profond des élus concernés, qui vivent dans la crainte permanente, non seulement d'accidents liés à la présence de loups jusque dans les villages et de chiens dans les chemins de randonnée, mais aussi d'accidents de chasse. Monsieur le ministre, il est nécessaire, à mes yeux, que chacun retrouve sa place. J'ai plaidé en faveur de la conservation d'une brigade loup je suis aujourd'hui convaincu qu'il faut soutenir les bergers et embaucher, si nécessaire dans le cadre de contrats aidés, des personnes dédiées à la sécurité. De plus, je crois nécessaire d'adapter la législation et, en particulier, les dispositions du code rural ayant pour objet la responsabilité des maires quant aux chiens de berger. À titre personnel, je suis enfin favorable à un autre mode de régulation de la présence lupine. Quiconque s'est trouvé face à un loup sait que le tir de prélèvement négocié n'est pas réaliste. Je plaide très clairement pour que le loup puisse- dans un cadre très réglementé, et lorsque la situation l'impose -être classé comme nuisible. Très bien ! Mes chers collègues, je souhaite vivement que cette proposition de résolution débouche sur des solutions pragmatiques, humaines et soucieuses de la préservation à court terme de nos territoires ! La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'être l'origine de la carte postale traditionnelle de la montagne, le pastoralisme est une activité économique. Il représente une agriculture vertueuse que pratiquent des femmes et des hommes passionnés, gardiens vigilants de l'équilibre entre la nature, l'homme et l'animal, et ce depuis des siècles. Je remercie les présidents Sophie Primas et Hervé Maurey, ainsi que nos collègues Patricia Morhet-Richaud, Jean-Noël Cardoux et Cyril Pellevat, d'avoir élaboré la présente proposition de résolution. à lancer l'alerte sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le pastoralisme et traduit le soutien de notre Haute Assemblée aux éleveurs sur cette question importante. importante. Il s'agit bien de préserver, au travers de produits reconnus, un maillon de la chaîne agroalimentaire dont les atouts touristiques et écologiques sont incontestables. L'entretien régulier de vastes étendues d'alpages par des troupeaux est indispensable à la lutte contre l'enfrichement comme à la protection contre les risques naturels.

Le pastoralisme est en cela un élément majeur de la protection et de la gestion des espaces naturels. Partout, les espaces pastoraux sont reconnus parmi ceux qui connaissent la biodiversité forte. Au coeur de nos parcs naturels, de nos réserves naturelles et de nos espaces protégés, ils constituent un enjeu de biodiversité majeur pour les écosystèmes. écosystèmes. Lors du comité interministériel de la biodiversité, le 4 juillet dernier, M. le Premier ministre a indiqué vouloir rémunérer les agriculteurs pour ce service qu'ils rendent à la nature. cette proposition de résolution vise à défendre une plus juste rémunération pour le pastoralisme qui tienne encore mieux compte des contraintes pesant sur cette forme d'agriculture. Ce serait une juste reconnaissance des contraintes spécifiques, liées aux conditions naturelles, à la saisonnalité et à l'isolement, auxquelles sont soumis les acteurs du pastoralisme. Évidemment, la question a été largement ouverte. Cette proposition de résolution met également en débat le soutien au retour de certains prédateurs, à l'image du loup ou, plus récemment, de l'ours, dont une nouvelle réintroduction dans les Pyrénées vient d'être annoncée. Si l'on peut concevoir aisément qu'il soit nécessaire de protéger des espèces relevant de la convention de Berne, la remise en cause de la viabilité économique d'exploitations agricoles en montagne ne saurait être la conséquence de cette protection.

Il me semble donc nécessaire qu'un arbitrage et un suivi fassent l'objet de discussions au sein de l'Union européenne. Il est tout aussi impératif que cette question trouve enfin, au sein du plan national au sein du plan national évoqué, des solutions pérennes offrant aux acteurs du pastoralisme toutes les sécurités nécessaires à la poursuite de leur activité économique. La compatibilité du pastoralisme avec la présence du loup est en question ; un équilibre doit donc être recherché, sans jamais perdre de vue que les acteurs du pastoralisme sont les pionniers de la biodiversité et des garants de la qualité. Le groupe Union Centriste votera donc en faveur de cette proposition de résolution.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite en premier lieu remercier nos collègues pour leur travail complet et ambitieux sur le pastoralisme.

Monsieur le ministre, il est certain que parler de loup, d'ours, de prédateurs et de pastoralisme au sein de notre hémicycle parisien peut faire sourire. Je me souviens encore du mépris d'un ancien ministre de l'agriculture lors d'une séance de questions d'actualité au Gouvernement- les agriculteurs n'ont pas oublié Nous savons par avance que nombre d'observateurs s'interrogeront sur l'utilité de notre démarche. Pour certains d'entre eux, le problème de l'articulation entre pastoralisme et prédateurs se résume à une ou deux brebis tuées par an ... Pourquoi donc débattre d'un tel sujet ? Mais cela est bien loin de la vérité ! Il est plus que jamais nécessaire et urgent de le rappeler et de porter ici, au coeur de notre représentation nationale, au Parlement, le cri de désespoir des éleveurs qui, chaque jour, pratiquent leur activité la boule au ventre. Oui, la défense du pastoralisme est d'une importance majeure ! Depuis des siècles, ces pratiques sont présentes en France ; elles façonnent le territoire et le protègent. Cependant, cette activité est aujourd'hui en danger. Avec plus de 12 000 attaques de loup par an, dont 40 % se déroulent désormais en plein jour et, parfois, à proximité des habitations, les bergers, mais également les élus locaux ne peuvent plus faire face. Avec un taux de croissance annuel de près de 20 %, près de 500 loups adultes seraient présents en France. Face à ces chiffres, le montant des indemnisations, plus que jamais nécessaires, explose, jusqu'à atteindre désormais plus de 20 millions d'euros par an. Dans le même temps, les inquiétudes sont toujours plus nombreuses sur le terrain.

Cela aboutit à des drames humains face auxquels les élus locaux n'ont pas de moyens de réponse. Aussi, certains d'entre eux décident de fermer l'accès aux chemins de randonnée pour éviter de subir de telles tragédies. L'activité économique du pastoralisme étant elle-même menacée, de nombreux éleveurs décident de mettre fin à leur activité. Cette situation démontre finalement trois choses : le loup gagne la bataille géographique, en avançant sur les terres le loup gagne la bataille économique, car la détresse des éleveurs est telle qu'ils sont nombreux à vouloir arrêter leur activité ; le loup, enfin, est en train de gagner la bataille politique face à l'absence de propositions des pouvoirs publics. Nous connaissons d'ores et déjà les réponses qui nous seront faites. La convention de Berne et la directive Habitats nous empêchent de mettre en place des politiques plus fermes sur le sujet. Mais peut-on encore considérer le loup comme une espèce en voie de disparition ? Monsieur le ministre, comment peut-on le prétendre, quand l'ambition du Gouvernement est de réformer et de faire avancer l'Europe ? La détermination de chacun devrait permettre de revenir sur ces textes, alors qu'une majorité de pays européens est désormais affectée par la question des prédateurs. Le Gouvernement aurait présenté un plan Loup 2018-2023 ambitieux. Toutefois, pour les éleveurs, les mesures prises ne paraissent pas à la hauteur face aux réalités du terrain et aux attentes des acteurs du pastoralisme. Ce plan illustre parfaitement le peu de considération qu'a le Gouvernement pour les territoires. Face à une telle indifférence, j'espère que la proposition de résolution que nous adopterons permettra au Gouvernement de réaliser des avancées, d'amender le plan Loup et d'ouvrir des négociations sur le sujet européen afin de revoir à la hausse le nombre de prélèvements par rapport au nombre de loups présents sur les territoires ; c'est une question de bon équilibre de la biodiversité. En conclusion, je citerai le Président de la République : le 25 janvier 2018, il annonçait vouloir remettre « l'éleveur au milieu de la montagne » ; or, aujourd'hui, nous constatons que ce sont toujours les loups qui sont au milieu de la bergerie

Vos nombreuses auditions d'élus locaux et d'éleveurs, ainsi que la diversité des acteurs impliqués, nous fournissent une matière bien précieuse pour continuer à travailler.

on estime à 430, en sortie d'hiver 2017-2018, le nombre de loups présents sur le territoire national, et ce dans plus de 74 zones de présence permanentes, dont 57 comprennent des meutes.

L'indemnisation est quant à elle assurée par le ministère de la transition écologique et solidaire, à hauteur de 3,5 millions d'euros par an. Bien sûr, ces montants ne couvrent qu'une partie des dépenses nécessaires à la cohabitation du loup et de l'élevage sur ces espaces d'agropastoralisme. La détresse et l'angoisse des éleveurs sont réelles et compréhensibles ; je veux particulièrement leur dire que l'État est à leurs côtés,

Ce plan, finalisé en février dernier, guidera l'action du Gouvernement sur les six prochaines années. Il offre plus de moyens aux éleveurs et les remet au centre de la montagne, tout en offrant au loup un cadre protecteur. -pourra être révisé une fois le seuil de viabilité de 500 loups atteint. On y est déjà ! Même si j'ai conscience de ses limites au regard des attentes des acteurs agricoles, ce plan comporte de réelles avancées. de réelles avancées. En effet, il inscrit le principe d'une gestion adaptée aux impacts sur l'élevage et aux réalités des territoires. En outre, l'État poursuit son appui financier au déploiement des mesures de protection des troupeaux en fonction de l'expansion du loup. Vous le savez, l'un des éléments clefs de cette protection est le gardiennage par l'activité des bergers. C'est pourquoi le Gouvernement s'engage à négocier avec la Commission européenne la prise en charge à 100 % du coût du berger salarié, contre 80 % dans le plan précédent. ailleurs, la prédation sera abordée dans la formation des bergers ; l'attractivité du métier sera renforcée et le recrutement ainsi facilité. Un réseau de référents techniques, déjà opérationnel, permettra de diffuser les savoir-faire et de sécuriser l'utilisation des chiens de protection, sous forme de formations collectives ou de conseils individuels. Par ailleurs, une expérimentation menée dans les parcs nationaux de la Vanoise et du Mercantour vise à mobiliser une brigade de bergers mobiles expérimentés pour venir en aide aux éleveurs dans les foyers d'attaque les plus importants. Au-delà de la protection des troupeaux, le soutien au pastoralisme constitue un élément très important de ce plan. Des plans de soutien à l'économie de montagne, sur le modèle pyrénéen, vont voir le jour sous la houlette des préfets coordonnateurs des Alpes et du Massif central. La conditionnalité de l'indemnisation des dommages, c'est-à-dire l'obligation, pour un éleveur souhaitant être indemnisé, d'avoir, au préalable, mis en place des moyens de protection suscite des incompréhensions, Cette obligation, qui résulte de l'application des lignes directrices agricoles européennes, vise à assurer la sécurité juridique et financière du dispositif d'indemnisation. d'indemnisation. Conscient des contraintes qu'il impose, le Gouvernement veillera à un déploiement progressif de ce principe. Par exemple, il ne s'appliquera ni aux nouvelles zones de présence du loup ni à la première attaque. Des dérogations seront possibles sur les fronts de colonisation où la mise en oeuvre de mesures de protection est difficile, ainsi que pour les troupeaux considérés comme non protégeables. Une concertation avec les représentants de la filière va définir des critères pertinents. Une usine à gaz ! Il n'y a là rien de « techno », ce sont des mesures simples et rapides à mettre en oeuvre. J'ajoute que la révision de ce régime d'indemnisation des dommages liés à la prédation intègre également une revalorisation des barèmes et la prise en compte des pertes indirectes telles que la baisse de lactation, ou encore le stress des animaux. Ces

Cette année, la destruction de 10 % de la population de loups, soit 43 animaux, a été autorisée. Ce taux pourra être porté à 12 % en cas de nécessité. De plus, pour protéger les troupeaux toute l'année, la nouvelle réglementation donne le droit aux éleveurs de continuer à pratiquer des tirs de défense au-delà du plafond annuel de loups pouvant être tués. Le plan prévoit également une libéralisation des modes de tir, notamment du tir de défense simple avec une arme à canon rayé, et un accès plus rapide au tir de défense renforcée. de procéder à des tirs d'effarouchement sans autorisation administrative est également accordée. Le renforcement des pouvoirs des préfets pour une gestion adaptative et de proximité améliorera l'efficacité de ce dispositif. Pour le suivi des populations de loups, il est indispensable de se fonder sur des données solides et des méthodes de collecte rigoureuses. Ce travail est mené par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, seul organisme en mesure de délivrer des informations fiables. Les données sur les constats de dommages sont disponibles sur la base de données Géoloup. Le plan Loup prévoit le regroupement de l'ensemble des informations dans une base de données nationale réactive, partagée et multifonctionnelle, qui comportera un suivi des dommages, des cartes, et un certain nombre de graphiques très utiles pour l'ensemble des éleveurs. Comme vous le savez, les engagements de la France en matière de préservation de l'espèce nous obligent à respecter l'objectif de viabilité de 500 loups. Une fois cet objectif atteint, il conviendra de revoir ensemble les modalités de gestion de l'espèce. Par ailleurs, un axe fort du plan Loup vise à adapter l'intervention publique à l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier pour l'amélioration des techniques de protection des élevages et d'effarouchement du loup. Des travaux seront menés avec l'appui du conseil scientifique permanent du plan. Ce conseil, en cours de mise en place, constituera une instance experte en matière d'éthologie, de systèmes agropastoraux, d'effets des tirs de loups sur la prédation et la population, ou encore de techniques d'effarouchement. Enfin, une étude prospective pluridisciplinaire sur le pastoralisme à l'horizon de 2035 est lancée afin de mieux mesurer la capacité du pastoralisme à se maintenir, voire à se développer en présence du loup. Ses conclusions auront vocation à éclairer les choix politiques futurs. futurs. Le plan Loup fait l'objet d'un suivi, d'informations et d'échanges dans le cadre du groupe national Loup, réuni trois fois l'an, présidé par le préfet coordonnateur et regroupant les acteurs concernés : organisations nationales socioprofessionnelles et associatives, administrations administrations et établissements publics. Cet espace de dialogue doit permettre un traitement équilibré du sujet au regard des différents enjeux. Ce plan ouvre une nouvelle page des relations du pastoralisme avec le loup, ce qui- je l'espère -permettra une cohabitation plus apaisée. Je comprends l'urgence, je comprends aussi les craintes. Alors, sachez que je serai particulièrement attentif à la mise en oeuvre rapide et efficace des actions prévues. Nous évaluerons d'ailleurs ce plan à mi-parcours, avant le déploiement de la deuxième phase, pour adapter si nécessaire ses actions. Comme pour le loup, le plan d'actions Ours brun 2018-2028 vise à concilier la présence de l'ours avec le pastoralisme et à diminuer la prédation sur le bétail. Des accompagnements sont également prévus. Vous avez été nombreux à en faire état. Nous faisons confiance aux acteurs et aux élus locaux pour dépassionner le débat et construire ensemble cette coexistence sur le long terme. Je terminerai mon propos par une note optimiste sur le pastoralisme, sans occulter pour autant les difficultés rencontrées sur nos territoires. Comme le souligne parfaitement votre proposition de résolution, le pastoralisme est une pratique ancestrale et collective qui a modelé profondément les milieux montagnards français et leurs paysages. Nous y sommes attachés, car des femmes et des hommes participent chaque jour à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité sauvage, la variété de la flore des prairies de montagne et de la faune associée, mais aussi à la conservation de la biodiversité domestique, de nos races de vaches et de brebis adaptées à ces milieux spécifiques et difficiles, une forme de biodiversité elle aussi à préserver et à mettre en valeur.

Ces femmes et ces hommes ont su tirer parti des contraintes du milieu naturel pour développer des filières remarquables et des produits de qualité qui font l'excellence du patrimoine gastronomique français et assurent à certaines filières sous signe de qualité des prix du litre de lait payés au producteur parmi les plus élevés de France. Certes, ces expériences ne sont pas reproductibles partout et des différences existent entre les territoires.

N'oublions pas les ressources et les capacités d'adaptation et d'innovation de ces territoires et de leurs habitants, sur lesquelles nous comptons pour redonner espoir à nos éleveurs Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation est pleinement mobilisé au quotidien pour accompagner les territoires et leurs filières, notamment les plans de filière qui sont nés des États généraux de l'alimentation. Je serai particulièrement attentif à la prise en compte des enjeux du pastoralisme et à son soutien dans le cadre de la PAC d'après 2020. Pour conclure, je ne peux que vous inviter vivement à poursuivre vos travaux et à inciter les acteurs concernés à participer à la mise en oeuvre et au suivi du plan sur le terrain. Cela, à mon sens, rend encore prématurée l'adoption de votre résolution. La discussion générale est

Nous ne pouvons que vous soutenir dans cette voie, qui est également celle que nous défendons. Toutefois, si nous approuvons le fond, nous nous interrogeons sur la méthode. Quelles que soient les priorités politiques, pouvons-nous continuer à loger tout le monde à la même enseigne ? Sénateur ultramarin, je suis toujours frappé par les velléités d'uniformisation de la métropole, et ce depuis de nombreuses années. Votre gouvernement a déjà évoqué l'encouragement à la différenciation. Laissons de l'air aux territoires. Laissons-les innover. Ils savent mieux que personne ce qui est bon pour leur population. J'en veux pour preuve deux exemples. exemple, c'est votre réforme de l'abattement fiscal pour les populations d'outre-mer, abattement pourtant essentiel pour les classes moyennes. Cette mesure permettait de compenser la vie chère, en partie liée à l'octroi de mer. Vous annoncez que les sommes économisées seront réallouées à l'outre-mer : je vous demande des assurances sur la pérennisation de ce dispositif. Le second exemple, c'est la suppression de la TVA non perçue récupérable. Ce dispositif a pourtant des effets positifs sur le financement des investissements productifs dans nos territoires d'outre-mer. Ces mesures ne sont pas des avantages indus. Elles sont le reflet des sujétions et des spécificités des outre-mer. Les supprimer ne supprime pas les différences ! Madame la ministre, dans ce budget et dans les budgets mieux respecter les différences entre les territoires, riches et pauvres, ruraux et urbains, métropolitains et ultramarins ? La parole est à Mme la ministre des outre-mer. Monsieur le sénateur, le Gouvernement a choisi de placer ce budget sous le signe de la transformation et du soutien aux projets dans les territoires. Vous avez raison, il faut garder cette différenciation et, pour cela, « donner de l'air »- je reprends vos propres termes -aux territoires, aux projets et aux solutions. Bien sûr, les dépenses fiscales que vous évoquez ne sont pas des avantages indus, mais

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'intérieur, qui n'est pas là. Où Depuis plusieurs semaines, on ne compte plus les boucheries, charcuteries, poissonneries et fromageries harcelées, attaquées, détériorées au nom d'une cause prétendument animale. Vendredi dernier, l'abattoir de Haut-Valromey, dans l'Ain, a été la cible d'un incendie criminel, laissant 80 employés au chômage technique. Les mêmes activistes tentent d'empêcher ou de perturber de nombreuses activités liées au monde rural, pourtant exercées légalement. Les associations à l'origine de ce vandalisme sont ultra-minoritaires, mais bénéficient de forts soutiens médiatiques et financiers. Personne ne conteste la nécessité de prendre en compte en compte le bien-être animal, aussi bien celui des animaux d'élevage que celui des animaux de compagnie, mais il n'est pas acceptable qu'une très faible minorité veuille imposer par la violence un mode de vie mettant en cause l'équilibre de notre société au nom d'une utopie importée des pays anglo-saxons. Si de telles actions perdurent, des affrontements sont à redouter. Que compte faire le Gouvernement pour mettre fin à de tels agissements et protéger dans notre société civilisée ceux qui exercent pacifiquement des activités légalement autorisées ?

jamais nous ne pourrons accepter que, au nom de cette liberté de choix, certains atteignent au principe même de la libre vente, de la libre exploitation, de la libre commercialisation et même de la sécurité,

il ne faut évidemment pas mettre tout le monde dans le même sac, mais certains comportements nécessitent une attention toute particulière. Dans le même esprit, le Gouvernement a reçu le président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs voilà quelques semaines, pour mettre en place des observations, des surveillances

Lorsque des exactions ont lieu, il faut que des investigations judiciaires soient systématiquement menées. Ainsi, les 10 et 11 septembre, des investigations diligentées par la sûreté de Lille conduit à l'interpellation de six activistes à l'origine de nombreuses dégradations. Sachez, monsieur le sénateur, que le Gouvernement restera totalement engagé et attentif pour qu'aucune situation ne dégénère.

du nouveau règlement européen qui exclut tous les ports français du corridor mer du Nord-Méditerranée pour le fret maritime reliant l'Irlande à l'Europe continentale. Jusqu'à présent, la majeure partie de ce trafic passait par les ports du Royaume-Uni. Dans la perspective du Brexit, la Commission européenne envisage le retour des barrières douanières dans les ports britanniques et anticipe ainsi la nécessité pour les Irlandais de remanier leurs itinéraires de fret maritime. Cette situation est pour nous une opportunité à saisir. Elle peut donner un nouvel élan aux ports français et, ainsi, renforcer leur attractivité. Si elle est maintenue, cette révision fera des ports du Benelux, comme Anvers ou Rotterdam, les grands gagnants du Brexit. vous concevez bien que cette décision serait inacceptable. En réponse aux interrogations formulées auprès de la commissaire européenne aux transports, celle-ci a déclaré que ce projet ne remettait pas en question les financements en cours sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, dit MIE 1. Mais qu'en sera-t-il pour le MIE qui prévoit d'allouer un financement de 30,6 milliards d'euros aux infrastructures de transports sur la période 2021-2027 ? Nous pouvons présager qu'une telle position ne ferait qu'accentuer l'écart de développement entre nos ports et ceux de nos voisins d'ici à 2020 et aurait automatiquement une influence sur les fléchages financiers du MIE 2. Cette hypothèse ne nous convient évidemment pas. C'est pourquoi, madame la ministre, nous aimerions connaître vos positions et propositions lors des négociations avec la Commission européenne, mais aussi les ports que vous souhaiteriez voir réintégrés au corridor, ainsi que la date d'entrée en vigueur de ce règlement. La parole

cette proposition de la Commission européenne n'était pas acceptable. J'ai eu l'occasion de le dire en ces termes à la commissaire européenne dès le mois d'août dernier. L'annonce prématurée de cette proposition était d'autant plus surprenante que nous avions d'ores et déjà engagé des échanges, notamment entre opérateurs français et irlandais. J'ai rencontré la commissaire européenne aux transports le 18 septembre dernier et je peux vous dire que notre mobilisation commence à porter ses fruits. J'ai défendu l'inscription de l'ensemble des ports français concernés dans ces nouveaux tracés. Il en ressort que les ports qui figuraient déjà dans le corridor mer du Nord-Méditerranée, notamment le port de Calais, y resteront. J'ai également sollicité, sans attendre la révision des corridors, la mise à disposition de moyens financiers exceptionnels par l'Union européenne pour tenir compte des effets du Brexit. Des discussions sont en cours sur ce sujet. Il est clair que les ports français doivent avoir toute leur place dans les nouvelles routes maritimes post-Brexit. C'est non seulement une évidence, mais c'est une conviction forte du Gouvernement que nous partageons avec tous les élus des territoires. Nos ports disposent d'atouts exceptionnels, et nous allons continuer à les défendre. C'est la raison pour laquelle, outre les débats au sein du Conseil et au Parlement, nous allons travailler étroitement avec l'Irlande sur ces sujets. Vous le voyez, la mobilisation du Gouvernement est totale. Vous pouvez compter sur ma détermination, comme je sais pouvoir compter sur votre soutien. La parole

de l'innovation. Permettez-moi de commencer mon propos en rendant hommage à un grand scientifique français, Gérard Mourou, qui vient de se voir décerner le prix Nobel de physique. Madame la ministre, la plateforme Parcoursup, mise en place en janvier 2018, répond à un objectif : recueillir et gérer les voeux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français. Ce nouveau dispositif est venu remplacer APB, un système très critiqué pour n'avoir pas su gérer l'afflux de demandes, ce qui avait conduit à instaurer le tirage au sort dans les filières en tension, véritable loterie, source d'injustice. syndicat représentatif des étudiants, a noté un enjeu essentiel dans cette réforme : réduire les disparités d'accès des étudiants aux filières qui leur correspondent et favoriser la mixité sociale. L'instauration d'un quota de mobilité, par exemple, a permis à 43 % des candidats de l'académie de Créteil de se voir acceptés à Paris, contre 26 % en 2017. Dans la phase principale toujours, 65 % des bacheliers professionnels ont reçu une proposition en section de technicien supérieur, contre 53 % en 2017. Moins de 1 000 bacheliers restent aujourd'hui en accompagnement. Me

Quelles mesures entendez-vous prendre dès l'année prochaine pour raccourcir les délais d'attente dont ont souffert certains élèves, engendrant un stress bien compréhensible

moins d'un an après l'annonce du plan Étudiants et à peine plus de six mois après la promulgation de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les trois engagements qui avaient été pris par le Premier ministre et moi-même ont été tenus. Ce n'est de n'affecter aucun étudiant par tirage au sort, de remettre de l'humain dans le système et de faire en sorte que la rentrée universitaire 2018 coûte moins cher que la rentrée universitaire 2017. Le bilan est clair, les chiffres sont là : nous sommes très loin des légendes urbaines qui ont circulé pendant l'été. Ce sont effectivement 23 % de boursiers

Les professeurs principaux, l'ensemble des équipes pédagogiques des établissements ont travaillé d'arrache-pied afin d'obtenir ces résultats ; c'est à eux que nous les devons. Parcoursup et la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants sont une réussite, c'est parce que l'immense majorité du corps enseignant soutenait l'idée qu'il était temps de changer les méthodes d'accès à l'enseignement supérieur.

Le 6 septembre dernier, M. Gilles Carrez, député du Val-de-Marne, remettait à M. le Premier ministre son rapport sur le financement du Grand Paris Express. À cette occasion, la presse a rapporté plusieurs pistes de travail à l'étude, notamment la hausse de la taxe sur les surfaces de bureaux, la hausse de la taxe de séjour et la hausse de la taxe Grand Paris. Madame la ministre, s'il n'est pas question de remettre en cause le bien-fondé du Grand Paris Express, il faut enfin être lucide sur ce projet pharaonique qui engloutira, durant plusieurs dizaines d'années, les investissements en transport de toute la région Île-de-France, au détriment de la modernisation du réseau existant qui est au bord de l'implosion. Pour rappel, ce projet, dont vous avez hérité, était initialement estimé à 26 milliards d'euros. Nous en sommes aujourd'hui à 35 milliards d'euros, et nous sommes nombreux à penser que la note va encore s'alourdir dans les années à venir. venir. Avec ses 200 kilomètres de tunnels, ce projet de transports a été conçu comme il y a trente ans, alors que d'autres solutions existaient et existent encore ; des solutions plus rapides à mettre en oeuvre, plus écologiques, plus adaptées aux bassins de vie et, surtout, beaucoup moins coûteuses. Par ailleurs, le compte n'y est pas pour les 5,5 millions d'habitants de la grande couronne ni pour les entreprises qui se battent pour se développer en périphérie de Paris et subissent la dégradation du réseau existant, notamment sur les lignes du RER. Il y a urgence. Nous ne pourrons pas attendre quinze ans de plus. Les accidents sur les voies se multiplient et des drames ont eu lieu récemment,

d'augmenter la taxe Grand Paris, ce qui aurait pour conséquence de continuer à faire payer aux habitants et aux entreprises de grande banlieue des infrastructures de transport qui se développent quasiment uniquement dans la zone dense ? La parole est à Mme la ministre chargée des transports.

transformer la vie de millions de Franciliens. C'est un projet d'une ampleur exceptionnelle, avec la construction de 200 kilomètres de lignes nouvelles, 68 gares. Le Grand Paris Express représente un défi absolument hors normes, mais qui doit bénéficier à l'ensemble des habitants d'Île-de-France, grâce notamment aux nombreuses gares d'interconnexion, ainsi qu'aux lignes de rabattement. Il ne faut pas opposer la réalisation du métro du Grand Paris et la modernisation, l'amélioration des réseaux existants. C'est tout le sens du plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France qui associe la région, les collectivités et l'État. Je rappelle que 7,6 milliards d'euros sont prévus dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020 au profit de projets et d'améliorations très concrètes pour les Franciliens, qu'il s'agisse du prolongement du RER E, des schémas directeurs des RER, dont le RER C que vous connaissez bien, des prolongements de lignes de métro ou de tramway, des lignes de tram-train, sans parler de l'effort exceptionnel sur la régénération ferroviaire. Je rappelle que nous allons consacrer 50 de financement de plus dans cette décennie que ce qui a été fait au cours des dix dernières années. C'est donc un programme extrêmement ambitieux, nécessaire, qui bénéficie à tous les territoires franciliens et qui est conforme à notre priorité : améliorer les déplacements du quotidien des Français pour donner à chacun la possibilité d'accéder aux emplois, aux services et à la formation. La parole

républicain citoyen et écologiste. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans le cadre des négociations sur le Brexit, la Commission européenne a choisi, par une décision autoritaire et technocratique, de redessiner les routes maritimes européennes. Si l'objectif est d'éviter l'isolement de l'Irlande en créant de nouveaux corridors, la solution retenue au coeur de l'été exclut les ports français de la façade nord, du Havre à Dunkerque. Nos ports faisaient déjà face à la « concurrence libre et non faussée » des ports belges et néerlandais, en particulier Anvers et Rotterdam, dont les moyens ne sont pas les mêmes- 900 millions d'euros de fonds européens pour Rotterdam contre 174 millions d'euros pour tous les ports français. Maintenant, la Commission change les règles, en bafouant elle-même le sacro-saint principe du libéralisme, en discriminant la France. Comme mes collègues de Seine-Maritime ou du Nord, je suis indignée par cette décision, qui aura évidemment des conséquences directes sur le port de Calais, pour lequel le commerce transmanche représente une part non négligeable du trafic. Nos ports, malgré les désengagements successifs de l'État, ont lancé toute une série d'investissements, 600 millions d'euros pour le seul port de Calais, visant également à la modernisation de leurs équipements, qu'il s'agisse du Havre ou ou de l'extension en cours du port de Dunkerque. Quel message pour les investisseurs, les salariés, les dockers et les industries ! Comment, madame la ministre, une telle décision a-t-elle pu être prise sans l'aval de la France et de son gouvernement ? Où en êtes-vous dans vos échanges avec la Commission ? Comptez-vous regarder passer les navires ou réagir ? La

Je le répète, cette proposition de la Commission européenne n'était pas acceptable- j'ai eu l'occasion de le dire à la commissaire lors de ma rencontre le 18 septembre dernier d'autant qu'elle fait fi de la réalité des trafics actuels, puisque la majorité des flux de marchandises entre l'Irlande et le continent passe aujourd'hui par le Royaume-Uni. L'analyse de la Commission fondée sur les échanges maritimes entre l'Irlande et la France ne peut donc pas préjuger les futurs échanges maritimes entre l'Irlande et le continent. J'ai donc défendu l'inscription de l'ensemble des ports concernés lors de ma rencontre avec la commissaire. Il en ressort d'ores et déjà que les ports qui figuraient dans le corridor mer du Nord-Méditerranée y resteront. Je le redis, Je le redis, les ports français doivent avoir toute leur place dans les nouvelles routes maritimes à l'issue du Brexit. C'est non seulement une évidence, mais une conviction forte du Gouvernement. de permettre à nos ports de tirer parti de tous leurs atouts. Nous allons nommer prochainement un coordinateur interministériel pour le Brexit qui pourra mener ce travail, en étroite liaison avec chaque port et les collectivités concernées. Nos ports disposent d'atouts essentiels pour ces échanges avec l'Irlande. Le port de Calais, comme vous l'avez rappelé, joue un rôle majeur dans les échanges entre le Royaume-Uni, la France et l'Europe. il faut vingt heures pour assurer la liaison entre Dublin et Cherbourg, contre trente-huit heures pour rallier Zeebruges. L'enjeu est donc clair : faire en sorte que l'ensemble des ports de la façade maritime soit bien intégré dans ces futurs échanges ; je pense à Calais, à Dunkerque ou au Havre, aux ports de l'axe Seine, mais aussi à Cherbourg, ainsi qu'aux ports bretons de Brest et Roscoff. La parole

exceptionnel du Calaisis. J'attends encore votre réponse à mon courrier. La parole

Vis-à-vis du pouvoir judiciaire, ensuite : les trois candidatures présentées pour la succession de François Molins ont toutes été écartées, en dépit d'un grand oral passé devant le Premier ministre. Ce rejet sonne comme une mauvaise manière faite à ces magistrats et comme un désaveu pour vous-même. Nous vous savons très préoccupée par le vaudeville de la place Beauvau et les portes qui claquent. Malgré tout, madame la garde pouvez-vous nous rassurer sur l'indépendance de la justice ? Pouvez-vous nous garantir la crédibilité du futur procureur de Paris ?

M. François Molins, que l'on puisse mettre en doute l'indépendance des procureurs en général, celle du procureur de Paris sur lequel vous m'interrogez en particulier. Et du suivant ? Qu'il s'agisse des commissions d'enquête créées par le Parlement comme des nominations des procureurs, il est toujours important de rappeler les principes constitutionnels. C'est ce que je voudrais faire en quelques mots, monsieur le sénateur. Le dialogue qui est naturellement entretenu entre la garde des sceaux, le Premier ministre et le Président de la République autour de la nomination d'un procureur important, celui de Paris, est un dialogue normal reposant sur un fondement constitutionnel, l'article 20 de la Constitution, qui précise que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Monsieur le sénateur Durain, quelle politique plus importante que la politique pénale de notre Nation ? Il est donc tout à fait naturel que les procureurs de la République soient situés sous mon autorité dans une chaîne hiérarchique et sous l'autorité du Premier ministre ; cela me semble tout à fait évident. Par ailleurs, la Constitution garantit également l'indépendance de ces magistrats, d'une part parce qu'ils sont libres de l'opportunité des poursuites, d'autre part parce que strictement aucune que strictement aucune instruction individuelle ne leur est adressée. Et mieux, même, le projet de révision constitutionnelle que j'espère avoir le plaisir prochain de porter devant vous conforte

Par ailleurs, nous souhaitons obtenir quelques garanties sur l'ambiance gouvernementale. Finalement, il y a ceux qui sont déjà partis- ils sont six -, ceux qui s'apprêtent à partir, font et défont leurs valises- y a-t-il encore un ministre de l'intérieur ? ? -, ceux qui regardent les prochaines municipales- quatre pour la seule ville de Paris ... Nous avons besoin d'un Gouvernement concentré sur ses tâches, au travail, où règne un peu d'ordre, d'un Gouvernement respectueux des autres pouvoirs, la justice et les parlementaires.

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Il y a quelques années, Roger Gicquel ouvrait son journal télévisé en déclarant : « La France a peur ». Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, les ruraux en ont ras-le-bol. Ras-le-bol d'être oubliés, ignorés et, plus grave, méprisés. La taxation du carburant atteint un niveau intolérable. Nos concitoyens vivant en montagne subissent donc une double peine entre la route et le coût du chauffage. Tributaires de leurs voitures, les ruraux sont donc les premiers ciblés par la limitation uniforme et aveugle de la vitesse à 80 kilomètres Dans les territoires, les cabinets des médecins généralistes ferment, aggravant les déserts médicaux ; et ne parlons pas des spécialistes ! Le sentiment d'enclavement n'est en rien diminué par l'internet, qui constitue une nouvelle fracture. Déjà privés d'un niveau acceptable de couverture mobile, les ruraux se voient aussi régulièrement privés de téléphonie fixe sur de longues périodes : qui s'en émeut ? Cette année, le Gouvernement a refusé de porter les pensions des agriculteurs retraités à 85 % du SMIC. Faire des cadeaux fiscaux aux super-riches et refuser une augmentation à ceux qui perçoivent 700 euros de retraite mensuelle est une bien curieuse manière de pratiquer la solidarité Les retraités ruraux, dans leur majorité, perdent du pouvoir d'achat. En effet, ayant pour nombre d'entre eux des revenus très faibles, ils sont déjà exonérés de la taxe d'habitation. La colère gronde dans les campagnes. L'élément déclencheur sera certainement la taxation du transport routier, souvent le seul moyen d'approvisionnement et d'exportation des productions locales. Après la révolte dans les urnes, nous verrons, je le crains, la révolte dans les champs. Les ruraux ne sont ni les premiers ni les derniers de cordée, mais les oubliés de la Macronie. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour redonner l'espoir aux millions de Français de la ruralité ?

nous devons éviter, les uns et les autres, une sorte de poujadisme rural. Nous avons aussi, et je le dis tel que je le pense, pour porter depuis longtemps ces dossiers,

Or ce monde, vous avez raison, considère qu'il est plus éloigné des centres de décisions qu'autrefois, qu'avant même la décentralisation. Cela, nous le vivons, et je dois dire que les fusions autoritaires de régions ou d'intercommunalités n'ont pas facilité les choses ... Je vous les choses ... Je vous le dis, au nom du Gouvernement, nous n'entendons pas changer une nouvelle fois les institutions. Nous entendons respecter les communes,

un sujet d'actualité puisque le Gouvernement finalise son projet de loi sur les mobilités et que sont enfin connues, après de nombreux mois d'attente, les conclusions de l'audit externe sur l'état de notre réseau routier national. Le constat, comme on pouvait s'y attendre, est sans appel. Il confirme la dégradation progressive de ce réseau, puisque, depuis 2007, le pourcentage de chaussées en bon état est passé de 57 % à 47 %, tandis que la proportion de chaussées nécessitant un entretien urgent, de surface ou de structure, a, elle, considérablement augmenté. Concernant les ouvrages d'art, si le rapport établit une relative stabilité du nombre de ponts en mauvais état, il alerte sur le volume croissant de ceux qui nécessitent un entretien. Dans ma région, 67 % du réseau routier non concédé mériteraient des travaux d'entretien.

Ces chiffres montrent la nécessité de réaliser un important effort d'investissements. Les tragiques événements de Gênes nous obligent à la plus grande vigilance en la matière et commandent une intervention affirmée de la part du Gouvernement. Notre commission de l'aménagement du territoire a d'ailleurs décidé la mise en place d'une mission d'information sur les ouvrages d'art. Le budget annoncé par le Gouvernement pour sa politique d'investissement, bien que considérable, reste malgré tout en deçà des attentes, notamment celles qui ont été formulées dans le cadre du les 13,4 milliards d'euros ne permettront pas d'atteindre le scénario 2, alors que, je le rappelle, le COI l'a bâti pour permettre la réalisation des ambitions affichées par le Président de la République. Je souhaiterais donc connaître, madame la ministre, les modalités de l'arbitrage ainsi réalisé, à la fois sur le montant global de l'enveloppe et sur les clés de répartition entre les différents secteurs de transports. La parole

Personne ne peut transiger avec cette exigence, qui ne doit plus être une variable d'ajustement, comme cela l'a été trop longtemps. C'est une priorité que je porte depuis mon arrivée à la tête du ministère, et c'est un choix que nous avons eu le courage de faire dès l'été 2017, le drame de Gênes nous ayant rappelé cet impératif. Mais nous n'avons pas perdu de temps pour agir et inverser la tendance à la dégradation de notre réseau routier. Dès 2018, nous avons augmenté de 100 millions d'euros le budget consacré à l'entretien et à la régénération des routes nationales. Nous avons aussi fait le choix de la transparence, en lançant des audits sur tous nos réseaux, notamment le réseau routier, audits qui ont été rendus publics en juillet dernier. J'ai également pris la décision de publier la liste des principaux ponts et leur état, car les citoyens ont le droit de savoir. Ce que cette liste nous montre, c'est que notre réseau n'est pas neuf et que nous avons des infrastructures qui vieillissent. Notre réseau fait toutefois l'objet d'un suivi extrêmement précis et rigoureux et, je tiens à le dire, il n'y a pas de situation d'urgence sur notre réseau. Quand des travaux sont nécessaires, ils sont entrepris. C'est notamment le cas sur le viaduc d'Echinghen que vous connaissez, sur lequel la SANEF est en train de réaliser des travaux. La programmation des investissements de transports portera cette ambition forte. Nous atteindrons un niveau jamais atteint : 850 millions d'euros d'ici à 2022, 930 millions d'euros sur le quinquennat suivant, à savoir 70 % de plus au cours de cette décennie que ce qui a été fait au cours des années précédentes. ces investissements supplémentaires représentent des besoins de financements supplémentaires. Nous devrons trouver des ressources pour financer ces besoins prioritaires, et je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour nous en donner les moyens. La parole

Quinze jours plus tard, il annonçait sa candidature à la mairie de Lyon, passant par pertes et profits son discours sur le nécessaire renouvellement de la classe politique. Puis l'on apprenait qu'il avait présenté sa démission au Président de la République, laquelle avait été Rebondissement aujourd'hui : on apprend qu'il maintient sa démission ... Un épisode comme celui-là, mettant en scène le Président de la République et l'un de ses ministres d'État, est inédit : nous vivons un grand moment politique Alors que l'insécurité en France atteint un niveau de moins en moins supportable pour la population, le Président de la République et le ministre de l'intérieur nous jouent une pièce de théâtre de boulevard on sort par une porte, on entre par une autre, et le suspense sur l'issue du spectacle demeure ... Lorsqu'on est élu, lorsqu'on est ministre de l'intérieur, on ne peut bien faire son travail que si l'on s'y consacre à 100

Avez-vous conscience, monsieur le Premier ministre, que les Français ne veulent plus de ces mises en scène, mais qu'ils attendent de la sincérité et des résultats ? Monsieur le Premier ministre, M. Collomb va-t-il oui ou non quitter le ministère de l'intérieur ?

nos choix en matière de réorganisation des services de renseignement, de coordination de l'action de ces services et d'augmentation des moyens budgétaires, matériels et humains mis à la disposition du ministère de l'intérieur.

de fonctions des membres du Gouvernement. Je prendrai donc mes responsabilités et j'aurai l'occasion de faire au Président de la République les propositions que les dispositions constitutionnelles prévoient et réservent au Premier ministre ! Le plus tôt

Il doit être clair pour tout le monde que personne ne souhaite contraindre un médecin à effectuer quelque acte que ce soit. C'est un principe général qui est garanti par l'article 47 du code de déontologie médicale.

Ce droit peine en outre à être effectif, 5 000 femmes se rendant encore chaque année à l'étranger pour une IVG. Cette double clause apparaît comme une double peine pour ces femmes. C'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion de Laurence Rossignol, nous proposons son abrogation. Madame la ministre, allez-vous enfin supprimer cette clause superfétatoire ? Surtout, quelles dispositions allez-vous prendre pour rendre effectif le droit à l'interruption volontaire de grossesse, par exemple en développant la place des sages-femmes et des médecins généralistes dans la pratique des IVG médicamenteuses comme instrumentales. Il s'agit, là encore, de garantir un droit que la loi reconnaît à toutes les femmes. La parole

d'évaluer les difficultés d'accès potentiel qui pourraient survenir dans certains établissements. Ce travail est en cours avec les agences régionales de santé. Vous pouvez compter sur mon plein et entier engagement

Il a déjà augmenté de 3 % la CSG payée par les retraités, il met en cause la pension de réversion des veuves et il va maintenant geler le niveau des retraites, ce qui entraînera, au fil de l'inflation, une perte considérable de pouvoir d'achat. Le président Macron prétend que les retraités sont des privilégiés. Il oublie que beaucoup de retraités ont commencé à travailler à 14 ans, qu'ils ont travaillé 40 heures par semaine, et qu'ils n'avaient que trois, puis quatre semaines de congés payés. Au contraire, les actifs d'aujourd'hui bénéficient du travail des générations précédentes. Ils ne commencent à travailler que très tard, ils font 35 heures par semaine, et ils ont cinq semaines de congés payés. Il faut donc être de mauvaise foi pour prétendre que les retraités vivent aux crochets des actifs. Les retraites ne sont pas des aides sociales ; elles sont le produit de cotisations versées tout au long d'une vie de travail. Face aux difficultés budgétaires que chacun connaît, il faut d'abord éviter de creuser les déficits par des mesures démagogiques telles que la suppression de la taxe d'habitation ou la baisse de moitié du prix du permis de chasse. Les retraités n'ont pas à servir de bouc émissaire pour boucher les trous. L'Allemagne, monsieur le ministre, vient d'augmenter les retraites de 3,4 %. N'est-il pas honteux que la France fasse exactement le contraire, en laminant le pouvoir d'achat des retraités ?

la réforme que nous avons annoncée, la diminution de la taxe d'habitation dès cette année compensera l'essentiel de l'augmentation de la CSG pour la plupart des retraités. Enfin, nous avons

en vingt secondes. Vos explications sont de la poudre aux yeux ! Je vais vous donner un exemple de mensonges que vous venez d'émettre.

conclure. Je conclus. Une étude économique vient de montrer qu'avec toutes ces mesures ciblées contre les personnes âgées, huit retraités sur dix

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi relative à la désignation aléatoire des comités de protection des personnes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

puisqu'elle vise à renforcer l'efficacité du tirage au sort des comités de protection des personnes, les CPP. Ce texte, auquel le Gouvernement, par la voix de Mme la ministre des solidarités et de la santé, était favorable à l'Assemblée nationale en première lecture, contribue à l'une des priorités du Gouvernement maintenir et renforcer l'attractivité de la France en matière de recherche impliquant la personne humaine tout en assurant la sécurité des personnes qui s'y prêtent. Cette mesure était également préconisée par le rapport sur les médicaments innovants, porté par les sénateurs Yves Daudigny, Catherine Deroche et Véronique Guillotin, que je veux ici remercier. Notre pays figure parmi les trois États européens les plus attractifs en matière de recherche, aux côtés de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Toutefois, depuis quelques années, les chiffres témoignent que nous accusons un retard pour les essais cliniques de phase 1, ceux qui correspondent le plus souvent à la première administration d'un médicament à l'homme. Aujourd'hui, nous devons non seulement rattraper ce retard pour tenir notre rang, mais aller au-delà, car notre pays a les capacités d'être un leader mondial de la recherche clinique. À l'occasion du 8 Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, qui s'est tenu en juillet dernier, le Premier ministre a souhaité que le renforcement de l'attractivité de la recherche française soit l'un des axes prioritaires. L'objectif est de faire de la France, à 5 ans, le premier pays européen en recherche clinique. Lors de son discours, le Premier ministre a bien noté que, ces dernières années, l'allongement des délais d'autorisation a entravé l'essor des essais cliniques, ce dont tout le monde pâtit la recherche, les patients et l'industrie. Aussi, il a annoncé vouloir réduire drastiquement les délais, en les abaissant dès 2019 à 45 jours pour l'Agence nationale de sécurité du médicament, et à 60 jours pour les comités de protection des personnes. Atteindre cet objectif suppose la mobilisation de chacun. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, a d'ores et déjà adapté son organisation en mettant en place une phase pilote de fonctionnement selon les exigences du règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments. Mais les promoteurs, les comités de protection des personnes, ou CPP, dont il est question aujourd'hui, La proposition de loi, qui a recueilli un accueil favorable de votre part lors de son examen en commission, apporte une solution à un point de cristallisation de la mise en oeuvre, en novembre 2016, de la réforme des recherches impliquant la personne humaine le dispositif d'attribution purement aléatoire par un système d'information du dossier de recherche à un CPP. Comme l'a déjà souligné Agnès Buzyn, ce texte permet de maintenir l'exigence de déontologie forte qui était légitimement voulue lors de la mise en place de ce tirage au sort, à savoir l'absence de tout conflit d'intérêts. Aussi, il s'agit bien d'améliorer le tirage au sort, mais certainement pas de le remettre en cause par un mécanisme qui reviendrait à une spécialisation des CPP. loi répond en même temps à la volonté des personnes malades et des professionnels de santé d'accéder dans les meilleurs délais, lorsque cela est possible, à des traitements innovants. Les travaux à l'Assemblée nationale ont ainsi conduit à ajouter de nouveaux critères afin de rendre le tirage au sort plus efficace. Le critère de disponibilité permettra de réguler plus finement l'attribution des dossiers et leur examen dans les délais prévus par la réglementation. Ce critère permettra de prévoir un nombre de dossiers traités par les CPP, afin d'éviter l'engorgement des comités, de lisser leur activité et donc d'éviter un retard dans l'examen des dossiers. Le critère de compétence, quant à lui, permettra de résoudre la question du défaut d'expertise de certains CPP pour l'examen de projets de recherche sur des thèmes particuliers. Les études avaient ainsi montré que des CPP rencontraient des difficultés à recourir à certaines expertises, les conduisant parfois à rendre des avis très au-delà des délais réglementaires. Le critère de compétence permettra à des CPP, compte tenu de leur composition et de leur capacité à recourir à l'expertise, de déclarer eux-mêmes, de façon transitoire, ne pas être en mesure d'évaluer certains types de dossiers. L'ensemble des CPP gardera bien une compétence générale pour donner un avis sur l'ensemble des dossiers de recherche. Cela ne ralentira pas les processus d'instruction, bien au contraire. Ces deux critères de « disponibilité » et de « compétence » contribueront à rendre plus efficient le tirage au sort. Ils sont à la fois nécessaires et suffisants pour répondre à l'enjeu de diminution drastique des délais d'autorisation des essais cliniques, dont chaque acteur pâtit, en premier lieu les patients. de loi intervient alors même qu'un ensemble d'actions visant à l'amélioration du fonctionnement des CPP est mis en oeuvre. En effet, le Gouvernement s'est engagé à améliorer les conditions d'exercice des CPP. Nous travaillons par ailleurs à la clarification de l'environnement réglementaire et à la qualification des recherches, ainsi que sur une grille commune d'évaluation des dossiers. Enfin, cette proposition de loi s'inscrit dans un cadre réglementaire européen en transition les règlements européens portant sur les essais cliniques de médicaments et sur les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic entreront en vigueur respectivement en 2020 et en 2022. Or, dans ce cadre, un CPP qui ne répondrait pas dans les délais prévus par ces règlements rendrait par défaut un avis favorable. Chacun pourra convenir un avis favorable. Chacun pourra convenir que cela serait préjudiciable à la sécurité des personnes se prêtant volontairement aux essais cliniques. Aussi, il est indispensable de permettre aux CPP de rendre des avis de qualité dans les délais.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a adopté le 25 septembre, en procédure de législation en commission, la proposition de loi relative à la désignation aléatoire des comités de protection des personnes. Dans un contexte où la concurrence internationale s'intensifie en matière d'implantation des essais cliniques, c'est le rang de la France dans la recherche clinique mondiale qui est en jeu. pays continue de faire partie des cinq pays accueillant le plus d'essais cliniques avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada, l'Espagne et la Belgique commencent à tirer leur épingle du jeu. Ce n'est toutefois pas par le seul prisme de l'attractivité que nous devons examiner les conditions d'évaluation scientifique et éthique des projets de recherche dans notre pays. La sécurité des volontaires doit demeurer notre première préoccupation, à l'heure où les esprits sont encore marqués par le souvenir de l'affaire Biotrial de 2016. L'indépendance et la pluridisciplinarité de l'évaluation éthique constituent l'ADN des CPP et c'est dans cette logique que notre commission a été à l'origine de l'introduction, dans la loi Jardé, du principe du tirage au sort des CPP. Le tirage au sort a-t-il allongé les délais d'examen des projets de recherche par les CPP ? Toutes les enquêtes recensées concluent à des délais moyens supérieurs à l'objectif de délai maximal de 60 jours, oscillant entre 70 et 85 jours. le tirage au sort a mis en lumière des inégalités entre nos trente-neuf CPP, qui préexistaient à ce mode de désignation. D'une part, certains CPP n'étaient pas préparés à traiter un flux continu de dossiers et ont dû ajuster leur mode d'organisation à moyens constants. D'autre part, plusieurs CPP rencontrent de véritables difficultés à mobiliser des spécialistes susceptibles d'éclairer le comité dans le domaine de recherche concerné. En 2017, trois CPP ne parvenaient pas à recruter de pédiatres, sept des experts d'essais de phase 1 et onze des experts en radioprotection. L'oncologie, l'oncohématologie, la virologie et l'ophtalmologie constituent d'autres spécialités pour lesquelles des CPP peinent à mobiliser des experts. Or, à partir de 2020 pour les essais cliniques de médicaments et 2022 pour les essais cliniques de dispositifs médicaux, le silence gardé au-delà des délais réglementaires vaudra accord, et non plus rejet. Il est parfaitement inconcevable que des projets de recherche puissent être entrepris sans validation éthique explicite. Il est d'ailleurs peu probable que les promoteurs s'y aventurent. On peut imaginer qu'ils se reporteront alors sur des pays plus réactifs que nous pour y organiser leurs essais. Il y va de l'accès des patients aux thérapies innovantes les essais cliniques suscitent un fort espoir chez des malades qui, après l'échec des thérapies traditionnelles, demeurent en attente d'un nouveau traitement, en particulier en oncologie et en oncohématologie, domaines dans lesquels se concentrent les essais de phase 1 en France. C'est pourquoi nos collègues Catherine Deroche, Véronique Guillotin et Yves Daudigny, dans leur rapport d'information sur l'accès précoce aux médicaments innovants, ont appelé au pragmatisme ils ont préconisé une modulation du tirage au sort selon la compétence afin d'attribuer un dossier de recherche à un CPP capable de mobiliser des experts dans le domaine concerné. La présente proposition de loi permet précisément de mettre en oeuvre cette recommandation, en modulant le tirage au sort des CPP selon leur disponibilité et leur compétence. L'attribution des dossiers de recherche tiendrait ainsi compte de la charge de travail du CPP et de sa capacité à mobiliser, en interne ou en externe, un spécialiste pertinent pour l'analyse du projet concerné. Au cours de l'examen de la proposition de loi en commission, Mme la ministre des solidarités et de la santé a confirmé que le critère de compétence serait apprécié souverainement par le CPP et que le système serait suffisamment évolutif pour tenir compte des nouvelles ressources en expertise identifiées par les CPP. À cet égard, nous plaidons pour la mise en place progressive par la commission nationale de la recherche impliquant la personne humaine d'un réseau national d'experts rapidement mobilisables et pour le déploiement d'un vaste programme de formation des membres de CPP et de leur secrétariat. L'objectif est que plus aucun CPP n'ait, à terme, à se déclarer incompétent sur une spécialité. Enfin, j'insiste sur l'impératif de prévention des conflits d'intérêts dans l'examen éthique des projets de recherche. Outre le tirage au sort et les déclarations publiques de liens d'intérêts auxquelles sont astreints les membres et experts des CPP, le fonctionnement collégial d'un comité, qui comporte des représentants tant du milieu médical que de la société civile, constitue une garantie puissante d'indépendance. Mes chers collègues, pour l'ensemble de ces raisons, notre commission a adopté sans modification la proposition de loi. J'invite donc le Sénat à adopter ce texte afin de permettre son application dans les meilleurs délais. La parole

Cette proposition cherche à orienter l'attribution d'un dossier de demande d'essais cliniques vers des comités de protection de personnes- CPP -« disponibles et disposant de la compétence nécessaire Les CPP sont chargés d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine. Ils se prononcent sur les conditions dans lesquelles le promoteur- celui qui prend l'initiative d'une recherche, par exemple le laboratoire -assure la protection des personnes, et notamment des participants, ainsi que sur le bien-fondé du projet de recherche, sa pertinence et sa qualité méthodologique. En bref, cette formation s'assure de la qualité éthique du projet de recherche. la randomisation- terme du jargon médical qui signifie tirage au sort -trouve sa source dans la loi Jardé de 2012. Ainsi, afin d'éviter les conflits d'intérêts, les promoteurs de recherches sur les personnes humaines ne pouvaient plus choisir les comités validant leurs projets.

Ce mécanisme, je cite, « réduit mécaniquement les risques de proximité entre le promoteur d'un projet de recherche et le CPP saisi de son évaluation éthique. » Le tirage au sort constitue un élément important de prévention des conflits d'intérêts. Toutefois, la situation et les délais actuels de traitement des dossiers par ces CPP peuvent apparaître préoccupants. En effet, comme le rappelait Mme la ministre des solidarités et de la santé, la moyenne de traitement des dossiers est actuellement de 71 jours, soit 15 jours de plus que les délais légaux, plus préoccupant que le nombre de dossiers examinés par les CPP s'accroît. Aussi, la proposition de loi vise à établir une répartition optimale de la charge de travail entre les C'est pourquoi le groupe La République En Marche, que je représente, défend la position de la commission, qui admet que la modulation de ce tirage au sort « au moins à titre transitoire » permettra de répondre au problème et de fluidifier le traitement des dossiers de recherche.

fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales. N'oublions toutefois pas que ce rapport préconisait aussi, je cite, « un renforcement du niveau d'expertise de tous les CPP par la mise en place de formations adaptées et d'un réseau d'experts rapidement mobilisables ». M. le rapporteur vient de le rappeler. Alors que les questions de bioéthique sont au coeur de l'actualité, nous avons ici l'opportunité d'améliorer de manière réelle et efficace la recherche médicale en France, en nous assurant que les spécialistes concernés pourront se prononcer plus rapidement sur sur des recherches qui, espérons-le, conduiront à des avancées thérapeutiques majeures. Mais il s'agit aussi de ne pas laisser se creuser un fossé entre l'industrie pharmaceutique française et celle d'autres pays, peut-être moins sensibilisés aux questions éthiques. La parole

qui sont bien souvent dans l'incapacité d'évaluer les projets de recherche dans le délai de 45 jours qui leur est imparti. Ils affirment que ces délais trop longs obligent les promoteurs à repousser la mise en oeuvre de leurs projets, parfois de plusieurs mois, ce qui nuit à la recherche médicale en France. Nous partageons ce constat : oui, les délais d'évaluation des projets sont parfois trop longs et oui, certains comités manquent d'experts compétents. Pour autant, la solution apportée est une fausse bonne idée, qui peut aggraver les défauts dénoncés, au lieu de les supprimer. Il ressort des auditions que les comités manquent de moyens humains et financiers. En effet, le budget qui leur est alloué stagne, voire diminue, alors que le nombre de dossiers à examiner est en croissance constante. En outre, En outre, l'accès aux experts est inégal, ce qui résulte non seulement de leur nombre restreint dans certains domaines complexes, mais également du manque d'attractivité, au sein des comités de protection des personnes, de la fonction de rapporteur, très faiblement indemnisée. Or la solution préconisée par cette proposition de loi n'est pas de donner aux comités les moyens nécessaires à l'exercice effectif de leurs missions, et notamment celle, centrale, de veiller à la protection des personnes qui se prêtent à une recherche médicale. La solution proposée consiste à réduire le nombre de comités parmi lesquels le tirage au sort est effectué. En réduisant ainsi la part de hasard, ne prend-on pas le risque de porter un coup à l'indépendance et à l'impartialité des comités ? En effet, le comité reconnu comme spécialiste de telle ou telle question pourra être facilement identifié. Cela ouvre la porte à de potentielles collusions entre lesdits comités et les promoteurs de projets, bien souvent des industriels, qui ont intérêt à ce que leur projet soit validé, et le plus vite possible, du fait d'enjeux financiers élevés. Par ailleurs, la mise en place de ce système ne présente aucune garantie démocratique. Mme la ministre des solidarités et de la santé nous a assuré, en commission, que la mise en relation entre les comités et les promoteurs des projets s'effectuerait au moyen d'un système informatique. Mais de simples algorithmes ne présentent pas des garanties suffisantes ! On ne sait pas comment ils sont développés, ni qui s'en servira. Enfin, Enfin, on ne sait pas quelles mesures seront prises pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts. Pour nous, la seule façon d'assurer le bon fonctionnement des comités et de garantir le respect de l'intégrité de la personne humaine est de donner des moyens financiers suffisants à ces comités, afin qu'ils puissent fonctionner de la façon la plus efficace possible. Vous dites vouloir renforcer l'attractivité de la France dans le domaine de la recherche, ce qui paraît légitime puisque la recherche concourt au progrès médical. Mais le secteur de la recherche est également un marché, dans lequel les entreprises sont en concurrence et cherchent à réduire les délais et les coûts. Pour cette raison, les exigences en la matière doivent être fortes. Or cette proposition de loi donne le sentiment de céder en priorité à des considérations économiques. Tout nous appelle aujourd'hui- je pense notamment aux différents scandales sanitaires qui ont, hélas, marqué l'actualité récente -à agir afin que les autorités publiques reprennent le contrôle sur les intérêts privés, en renforçant les moyens et les pouvoirs des comités de protection des personnes, mais également des autres organes publics amenés à intervenir sur les questions de santé. Nous le savons toutes et tous ici : le marché du médicament est une source considérable de profits, avec un chiffre d'affaires dépassant 1 000 milliards d'euros au plan mondial ! Nous ne pouvons laisser cette logique marchande prendre le pas sur la satisfaction des besoins de santé publique. C'est une question fondamentale liée à la maîtrise publique et à la transparence de la recherche médicale. Pensez-vous réellement que ce soit le rôle de l'industrie pharmaceutique de financer la recherche, de se charger de l'information médicale ou encore de la formation continue des médecins ? N'est-il pas temps, madame la secrétaire d'État, de donner aux pouvoirs publics un outil qui permettrait de sortir la chaîne du médicament de la loi du marché, ce qui passe, outre la production et la distribution des médicaments, par le développement de la recherche publique ? C'est tout le sens de notre proposition de pôle public du médicament en France

désignés par tirage au sort et dont l'avis positif est indispensable à la réalisation d'un projet de recherche impliquant des personnes humaines. Si le consensus est sans équivoque quant aux difficultés auxquelles font face les CPP, les moyens d'y remédier divergent et ne portent pas en leur sein les mêmes répercussions.

que leurs membres sont bénévoles, il leur est donc difficile de consacrer plus d'une journée par mois à l'étude des projets. La réponse la plus rapide et efficace à ces enjeux est-elle de nature législative ? Le doute est d'autant plus permis que l'auteur de la proposition de loi lui-même ne se cache pas de dire qu'elle n'a pas vocation à résoudre l'ensemble des problèmes ... Et nous ne sommes pas seulement dubitatifs quant aux supposées améliorations concrètes que permettrait la modification législative, car la liste des zones d'ombre est importante et les éléments de réponse apportés en commission n'ont pas permis de les dissiper. En premier lieu, nos doutes portent sur l'opportunité, y compris sur le plan temporel, de toucher par voie de proposition de loi, donc sans étude impact, au corpus législatif issu de la loi Jardé, fruit de longs débats parlementaires en 2012, et ce alors que nous serons saisis dans les prochains mois d'une loi de bioéthique, de bioéthique, qui aurait sans nul doute constitué un cadre approprié pour débattre, en connaissance, de l'ensemble des éléments et peser le poids de la nécessité et des implications de cette modification législative. lieu, pourquoi modifier la loi à l'approche de l'entrée en vigueur, au plus tard courant 2020, du règlement européen sur les essais cliniques de médicaments, qui instaurera de fait un cadre exigeant en matière de délais de traitement des dossiers ? Ce cadre sera non seulement à même de satisfaire les calendriers contraints des promoteurs de recherches, académiques comme privés, mais permettra également de sortir d'une logique de compétition entre pays européens au profit de la compétitivité européenne au niveau mondial. En France, les acteurs concernés n'ont d'ailleurs pas attendu l'entrée en vigueur de ce nouveau cadre pour se préparer à ses nouvelles exigences en matière de délai : nous avons en effet été le premier pays à lancer une phase pilote de deux ans afin de simuler le futur cadre et ainsi travailler sur la réduction des délais d'évaluation.

L'Agence s'est même fixé pour objectif d'instruire la moitié des demandes selon les futures exigences européennes sur l'année 2018, illustrant ainsi que les efforts à consentir sont essentiellement de nature organisationnelle et financière. Nos préoccupations ont également trait aux implications de la proposition de loi, qui introduit une pondération du caractère aléatoire de la désignation des CPP selon deux critères : la disponibilité et la compétence pour évaluer un projet de recherche. Premièrement, les modifications proposées renvoient à la mise en oeuvre- l'opérationnalité du principe de désignation aléatoire -et relèvent par conséquent davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif.

contre les potentiels conflits d'intérêts. L'article renvoie ainsi la détermination des conditions de la désignation aléatoire à un autre article, le L. 1123-14, qui dispose quant à lui que ces conditions sont fixées par un décret en Conseil d'État. Je pense que nous trouverions tous ici de bon sens que la partie réglementaire du code prévoie que le tirage au sort se fasse parmi les 39 CPP, dont le plan de charge permet l'étude d'un dossier dans les délais impartis, mais c'est bien le Gouvernement qui est habilité sur ce point, il n'y a nul besoin de toucher à la loi L'introduction du critère de compétence dans l'article L. 1123-6 est potentiellement plus problématique et nous ne disposons pas d'éléments sur la traduction concrète d'une telle modification. Comment s'assurer que suffisamment de CPP se déclarent compétents sur une aire thérapeutique ? Devrions-nous déterminer un seuil minimal de candidats pour sécuriser le caractère aléatoire de la désignation ? Et comment fixer ce seuil ? Ces questions laissent à penser que l'enjeu ne réside pas dans les compétences parmi les membres permanents des CPP, mais bien dans la manière dont ces derniers pourraient, par un dispositif souple et réactif, tel qu'un réseau de spécialistes agréés, accéder rapidement à l'expertise nécessaire. Une piste tout à fait prometteuse, soutenue par les associations de patients, est la constitution d'une liste d'experts à laquelle les CPP pourraient se référer.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 6 juin dernier, je prenais la parole à cette même tribune pour apporter mon soutien à la proposition de loi du président Milon autorisant les analyses génétiques sur personnes décédées. Cette proposition de loi a un point commun avec celle que nous examinons aujourd'hui : elles portent toutes les deux l'ambition d'une politique de santé plus efficiente en termes de prise en charge précoce et d'accès à l'innovation. Je ne peux que me réjouir, cette fois-ci, du soutien du Gouvernement. Dans son discours devant le Conseil stratégique des industries de santé, le 10 juillet, le Premier ministre a en effet présenté des mesures relatives aux essais cliniques, notamment la réduction du délai de réponse des CPP à moins de 60 jours. Un tel engagement est à saluer. En effet, l'innovation en santé est une chance, une opportunité majeure pour les patients atteints de maladies chroniques et graves, notamment dans le domaine de l'oncologie, mais comme cela a été rappelé, c'est aussi un atout pour la vitalité économique et le rayonnement de notre pays. Car il y a effectivement, en France, une économie de la recherche qui se porte bien, mais qui peine à conserver sa place parmi les leaders mondiaux. Face aux concurrents émergents, les trois pays les plus attractifs d'Europe- la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France -doivent être en capacité d'adapter leurs procédures au nouveau contexte international. Dans notre pays, l'innovation s'appuie depuis de très nombreuses années sur une exigence éthique, qui doit absolument être préservée. Certains ont pu émettre des craintes quant à d'éventuelles conséquences de cette proposition de loi. loi. Pour ma part, j'ai la conviction que l'équilibre entre exigence éthique et adaptabilité du système permettra de garantir son efficience. J'ai surtout la conviction qu'il faut agir. Avec mes collègues Catherine Deroche et Yves Daudigny, nous avons rédigé un rapport sur l'accès précoce aux médicaments innovants, dans lequel nous rappelions que l'accélération des innovations pose de nouvelles problématiques en matière de rapidité et d'équité d'accès à ces traitements. Pour certains patients, il peut tout simplement s'agir d'une question de vie ou de mort. Bien conscients du caractère prioritaire de l'expertise en matière d'essais cliniques, nous avions formulé, dans ce rapport, dix-huit propositions, dont celle de conforter les essais cliniques comme voie d'accès précoce aux traitements innovants, en renforçant notamment les CPP et leur expertise. Nous avons donc proposé d'adapter le système de tirage au sort, en prévoyant que celui-ci s'applique à un groupe restreint de CPP spécialisés, en fonction du domaine concerné par l'essai clinique. Depuis 2016, l'attribution des projets de recherche aux différents CPP s'effectue par tirage au sort simple. Nous sommes tous d'accord pour considérer ce tirage au sort comme nécessaire face aux conflits d'intérêts. Cependant, il nous faut également en mesurer les limites, notamment l'allongement des délais d'évaluation. Désignés de manière aléatoire pour l'examen d'un projet de recherche sur lequel ils n'ont pas les compétences en interne, certains CPP font appel à des avis extérieurs, ce qui allonge naturellement le délai d'évaluation. La composition des trente-neuf CPP n'étant pas homogène sur tout le territoire, il nous paraît nécessaire d'adapter ce tirage au sort pour qu'il s'applique effectivement à un groupe de comités disposant du niveau d'expertise requis pour chaque essai clinique. Il s'agit d'une question de bon sens, qui ne remet en cause ni l'exigence éthique ni la sécurité des patients. Il s'agit notamment de s'adapter au droit européen, qui nous mettra face à nos dysfonctionnements dès 2020, en entraînant par défaut un avis favorable des CPP ne répondant pas dans les délais prévus. Sans adaptation de notre système, cette réglementation européenne fait peser un risque sur la sécurité des personnes, un risque qui nous force à agir. Dans le même temps, il est nécessaire d'accroître le niveau d'expertise de tous les CPP grâce à des formations et à un réseau d'experts rapidement mobilisables. Comme notre rapporteur, j'insiste sur la nécessaire montée en compétences de l'ensemble des CPP. La liste de leurs expertises ne doit pas rester figée dans le temps, sous peine de voir ressurgir les risques de conflits d'intérêts. Dans notre rapport, nous avons également souligné l'importance de l'harmonisation des procédures d'évaluation et bien entendu du renforcement des moyens administratifs des comités. Sur ces différents points, nous resterons attentifs aux mesures concrètes qui seront proposées sur le terrain. de loi laissent au Gouvernement le soin de s'engager sur les moyens alloués aux CPP, ils apportent un début de réponse à la fragilisation de notre modèle. L'engagement du Gouvernement à faire appliquer cette disposition dans les meilleurs délais nous pousse à l'optimisme. Gageons que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et la nouvelle transformation de notre système de santé feront montre d'une même ambition en termes d'accès précoce aux innovations ! Dans cette attente, le groupe du RDSE votera en faveur de la proposition de loi.

nous sommes saisis de l'examen de la proposition de loi relative à la désignation aléatoire des comités de protection des personnes. Examiné selon la procédure de législation en commission, ce texte n'a fait l'objet d'aucun amendement. Les comités de protection des personnes ont pour mission d'analyser les projets de recherche impliquant la personne humaine. Ils déterminent si les protocoles envisagés sont de nature à préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants. À cette dimension éthique s'ajoute une mission scientifique d'évaluation de la méthodologie et de la pertinence de la recherche envisagée.

en France des projets de recherche les plus innovants. Ce sera le cas au moment de l'application du règlement européen qui s'y rapporte et qui permettra au promoteur de choisir l'État membre rapporteur sur son projet de recherche. Dans le même temps, le Gouvernement souhaite le renforcement de l'attractivité de la recherche clinique française. Il veut d'ailleurs en faire l'un des axes prioritaires du 8 Conseil stratégique des industries de santé.

Pour autant, le manque de moyens est patent. Certains CPP ont, effectivement, une charge de travail trop lourde et ne peuvent tenir les délais réglementaires. Par Par exemple, le secrétariat des CPP est souvent assuré par un seul équivalent temps plein et les périodes de congés et les arrêts maladie sont susceptibles de paralyser leur fonctionnement. En outre, depuis la mise en place de la procédure du tirage au sort, les projets peuvent être adressés à des CPP ne disposant pas d'experts nécessaires à leur examen. Notre rapporteur a noté que le concours d'experts spécialistes du champ de recherche est limité par la faible attractivité de cette fonction, indemnisée à hauteur de 67 euros pour toutes ces raisons, une revalorisation du programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé » correspondrait à l'objectif visé par le Gouvernement. J'ajoute que le niveau d'expertise élevé que requièrent des projets toujours plus à la pointe épuise par voie de conséquence le vivier des spécialistes. Enfin, la procédure actuelle ne permet pas ne permet pas aux CPP de se dessaisir une fois que le tirage au sort est effectué. Ainsi, même s'il est incapable techniquement de procéder à l'examen du projet, la seule issue pour le CPP est d'attendre l'extinction du délai réglementaire. Il le fait alors sans prononcer d'avis, ce qui équivaut à un rejet. Dès lors, cela relance un tirage au sort pour obtenir l'avis d'un CPP compétent. Ces lenteurs Ces lenteurs clairement identifiées finiront par disqualifier la France en la matière. L'article unique de cette proposition de loi vise à s'assurer que le tirage au sort attribue un projet à un CPP disponible et compétent. Ce principe ne remet pas en cause la prévention des risques de proximité entre le promoteur d'un projet de recherche et le CPP saisi de son évaluation éthique. Cette proposition de loi est susceptible de réduire le temps de traitement de l'examen des projets et elle mérite d'être soutenue. Il est toutefois urgent de doter les CPP d'aides financières et d'un appui administratif plus adéquat. Vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'État, le groupe Union Centriste considère que ce dispositif est un levier, mais qui devra être complété. C'est pourquoi j'appelle votre attention sur les recommandations faites par M. le rapporteur, tout en vous confirmant le vote favorable de notre groupe. La

monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre assemblée se penche aujourd'hui sur la question du régime législatif des recherches impliquant la personne humaine. La loi Jardé du 5 mars 2012 a apporté des améliorations significatives à ce régime en créant une catégorie unique de recherche et trois sous-catégories de recherche. Toute expérimentation ou tout essai organisé et pratiqué sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales est donc aujourd'hui encadré par la loi. Dans le fonctionnement de ce régime, les comités de protection des personnes, dits CPP, ont un rôle essentiel. Ils sont en effet chargés d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine au regard des critères définis dans le code de la santé publique. Ils se prononcent donc sur les conditions dans lesquelles le promoteur de la recherche assure la protection des personnes impliquées, notamment des participants, ainsi que sur le bien-fondé, la pertinence du projet de recherche et sur sa qualité méthodologique. Ces CPP sont aujourd'hui agréés par le ministère de la santé pour une durée de six ans, avec une compétence régionale. Afin d'assurer leur efficience et leur transparence, de manière pluridisciplinaire, avec 14 membres titulaires et 14 membres suppléants, répartis sur deux collèges et exerçant leurs fonctions de manière bénévole. Il convient d'ailleurs de rappeler, pour le saluer, le fait que ces personnes sont toutes soumises à l'obligation de déclaration publique d'intérêts afin que nul ne puisse contester la décision de ces comités. Cet édifice juridique est cependant biaisé. En effet, la composition des CPP est très variable d'un territoire à l'autre, au point que certains de ces comités ne peuvent pas garantir l'expertise nécessaire à l'évaluation des projets de recherche. En effet, la mécanique du tirage au sort a conduit à la nomination de CPP dont aucun membre ne disposait de l'expertise suffisante pour l'examen d'un projet de recherche dont il était saisi.

le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi de bon sens. La

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier notre groupe et son président, Bruno Retailleau, d'avoir demandé l'inscription, dans l'espace qui lui est réservé, de cette proposition de loi votée à l'Assemblée nationale en mai dernier. En effet, il est indispensable de renforcer l'efficacité du tirage au sort des comités de protection des personnes institué par la loi dite Jardé.

Notre attention a été attirée sur les difficultés rencontrées par les CPP pour accomplir leur mission, les 39 CPP présentant un niveau d'expertise et de réactivité inégal, voire insuffisant, en dépit de l'engagement bénévole et du dévouement de leurs membres manque d'expertise pour les essais particulièrement complexes, en particulier ceux qui sont spécifiques aux cancers, devenus extrêmement techniques ; forte hétérogénéité des niveaux et des pratiques ; dysfonctionnements administratifs liés à un manque de moyens. Notre proposition n° 16 vise à renforcer ces CPP et leur expertise en adaptant le tirage au sort en fonction du domaine de l'essai, en mettant en place des formations adaptées et à disposition des experts si besoin, en poursuivant l'harmonisation des procédures d'évaluation et et en renforçant les moyens administratifs. La France dispose de scientifiques de haut niveau, d'établissements d'excellence et de prises en charge de qualité. Néanmoins, on ne saurait nier une perte de vitesse de notre pays, des inégalités territoriales et, surtout, l'effet de cliquet que peut engendrer la réalisation d'un essai de phase 1 dans un autre pays que la France sur les phases suivantes. La proposition de loi que notre commission a examinée en procédure de législation en commission la semaine passée répond à ces difficultés en mettant en place ces deux critères d'attribution d'un dossier à un CPP : la disponibilité et la compétence. Je salue le travail de notre rapporteur, Jean Sol, qui a dressé un tableau pragmatique de la situation actuelle, mais aussi posé des exigences pour l'avenir. La ministre Mme Agnès Buzyn a pris des engagements forts ; nous serons vigilants sur la suite qui y sera donnée. Si le tirage au sort des CPP n'est effectif que depuis novembre 2016, les équipes de recherche clinique d'excellence s'en inquiétaient bien avant. En septembre 2015, le service des essais cliniques de Gustave-Roussy s'en était fait l'écho auprès du président Larcher lors de sa visite à Villejuif. En tant que présidente du groupe « cancer », créé en juin 2016, j'avais, dès juillet 2016, relayé auprès de Mme Marisol Touraine, alors ministre de la santé, les inquiétudes du département de recherche clinique de Gustave-Roussy et de son directeur sur le projet de décret d'application de la loi Jardé et ses conséquences sur les essais de phase 1 en oncologie pédiatrique, dont la méthodologie est très innovante. savoir que l'essai AcSé-ESMART aurait subi un retard majeur, voire un refus, avec la procédure actuelle de tirage au sort d'un CPP n'ayant jamais évalué un tel essai de médecine de précision. Je soutenais à l'époque la proposition d'un tirage au sort parmi un nombre de CPP limité pour les essais cliniques complexes en cancérologie, afin d'avoir un système d'autorisation fluide et efficace. C'est resté lettre morte, mais, aujourd'hui, grâce au vote conforme proposé en commission législative, un frein va être levé. Chercheurs, équipes soignantes, patients et familles de patients, laboratoires et biotechs l'attendaient. J'espère, madame la secrétaire d'État, que les délais réglementaires et opérationnels seront très courts- plus courts que ceux de la loi Jardé. Lors du Comité stratégique des industries de santé- CSIS -de juillet dernier, le Premier ministre s'est engagé à faire de la France le premier pays européen de recherche clinique en cinq ans. À l'heure où débute l'examen du PLFSS et du PLF 2019, nous serons attentifs sur ce que prévoit le Gouvernement sur ce sujet majeur. L'accélération des innovations est inouïe, notamment avec de nouvelles thérapies immunothérapie, médecine personnalisée -permettant d'améliorer les taux de survie de patients atteints de cancers ou de maladies rares, ainsi que leur qualité de vie. Soutenir l'innovation est un devoir dans un contexte budgétaire contraint, mais l'équilibre est délicat entre l'impératif de sécurité et le défi de la soutenabilité financière de notre système d'assurance maladie. Dans notre rapport d'information figurent cinq axes de propositions. Un premier pas est fait aujourd'hui, et j'aurai une pensée particulière notamment pour les équipes de chercheurs et les associations qui étaient attachées à cette évolution. La route est encore longue, mais ils peuvent compter sur notre mobilisation. Nous formons le voeu que le Gouvernement accompagne cette route

Les Républicains. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur du débat disposera d'un temps de parole de huit minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, trois ans après l'adoption de la loi Transition énergétique, et quelques semaines avant la présentation de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, ou PPE, il a paru essentiel au groupe Les Républicains de revenir, à l'occasion de ce débat, sur les grandes orientations de notre politique énergétique. Ce temps démocratique est d'autant plus nécessaire que le Parlement n'est aujourd'hui pas associé à la déclinaison des grands objectifs dans la PPE, malgré les sommes considérables qu'elle engage, qui justifieraient pleinement la discussion régulière d'une véritable loi de programmation, comme le réclame à raison notre collègue Jean-François Husson. Un tel débat permettrait d'ailleurs de remettre un peu de cohérence et de lisibilité dans une politique dont on dissémine les mesures au gré des projets de loi, le plus souvent sans lien avec leur objet ces derniers mois, on aura discuté des éoliennes en mer dans la loi « droit à l'erreur », du droit à l'injection du biogaz dans la loi ÉGALIM- on y reviendra encore dans la loi Mobilités -, ou encore de la suppression des tarifs réglementés dans la loi PACTE. Ce n'est ni sérieux ni à la hauteur des enjeux

au mieux irréalistes, au pire néfastes pour certains d'entre eux. Sur ces deux années, notre taux d'indépendance énergétique aura baissé de trois points du fait de la moindre disponibilité de nos centrales nucléaires, ce qui a contribué, avec la hausse des cours internationaux, à un rebond de 23 % de la facture énergétique française l'année dernière. En 2017, la consommation énergétique finale a aussi progressé de près de 1 grâce à la croissance économique, ce dont on ne peut que se réjouir, mais je rappelle que la loi visait une division par deux en 2050 Et dans le même temps, en raison du recours accru aux centrales thermiques pour compenser la baisse du nucléaire, les émissions de CO2 du secteur énergétique ont augmenté en 2017 de 4 % à climat constant, ce qui est une première depuis le milieu des années 2000. En nous donnant un avant-goût des effets d'une réduction trop brutale de la part du nucléaire, ces données démontrent que le Sénat avait eu raison de plaider pour une diversification plus progressive du mix électrique. du mix électrique. On regrettera qu'il ait fallu plus de deux ans au Gouvernement pour admettre que la date de 2025 n'était pas tenable, sauf à augmenter nos émissions Si nous sommes favorables au maintien d'un socle fort de nucléaire dans notre mix électrique,

et du mix électrique le moins carboné derrière la Suède, tout en assurant notre sécurité d'approvisionnement. Ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui avec l'essor des énergies renouvelables. Même ses adversaires, comme votre prédécesseur, monsieur le ministre l'ont reconnu : le nucléaire a l'immense avantage de faciliter la transition vers un mix énergétique plus renouvelable sans qu'il faille recourir à des moyens thermiques pour compenser l'intermittence de certaines énergies renouvelables, ni mettre en péril notre indépendance énergétique. Il est temps, comme nous l'avions plaidé à l'époque, de remettre de la raison dans ce débat où les passions aveuglent et font perdre le sens des réalités : qu'on le veuille ou non, la lutte contre le réchauffement climatique, qui est notre priorité, passe, aussi, par le nucléaire. Or, depuis l'annonce de l'abandon de la date de 2025, la ligne gouvernementale est floue : on nous parle tantôt de 2035, tantôt de 2030 ; on ne sait pas si la loi de 2015 sera modifiée, et, si oui, quand ; nous savons encore moins ce que contiendra la alors que la précédente avait tout simplement ignoré le sujet. Monsieur le ministre d'État, vous engagez-vous à ce que la PPE comporte le nombre, voire le nom des réacteurs à fermer et leur calendrier de fermeture ? Qu'adviendra-t-il ensuite ? Là encore, on ne sait pas où l'on va : un rapport d'experts commandé par le Gouvernement a récemment préconisé la création de six EPR à partir de 2025 pour assurer la relève et maintenir les compétences industrielles. Quelles suites y donnerez-vous ? Remettre de la raison, c'est aussi rappeler que le « tout-nucléaire » est un mythe, car le nucléaire n'a jamais représenté, au mieux, que les trois quarts d'une énergie, l'électricité, qui ne couvre elle-même qu'un quart de notre consommation énergétique finale, dont, je le rappelle, les deux tiers sont en réalité couverts par les énergies fossiles. C'est pourquoi nous pensons qu'au lieu de s'arc-bouter sur le nucléaire il vaut mieux s'engager résolument pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, ce qui sera bon non seulement pour la planète, mais aussi pour notre balance commerciale. Or, sur cette question, monsieur le ministre d'État, nous partageons le même objectif, mais nous ne prônons définitivement pas la même méthode. Là où nous souhaitons donner des solutions aux Français, vous leur donnez de nouveaux impôts ; là où nous voulons orienter les comportements, y compris par l'outil fiscal, vous voulez les contraindre, alors que nos concitoyens, en particulier dans les campagnes, n'ont souvent pas d'autre choix que de prendre leur voiture diesel pour aller travailler, ou de remplir leur cuve à fioul pour se chauffer. Votre gouvernement a pourtant décidé de les assommer avec une fiscalité énergétique qui explose sous l'effet de la taxe carbone et d'une convergence des tarifs de l'essence et du diesel qui fonctionne uniquement à la hausse. L'an dernier, nous avions calculé qu'entre 2018 et 2022 la pression fiscale augmenterait en cumulé de 46 milliards d'euros par le seul effet de la fiscalité énergétique. Vous aurez beau expliquer que la hausse sera compensée par ailleurs, les Français le constatent : le compte n'y est pas Vous dites vouloir une fiscalité écologique qui soit incitative et non punitive, mais le Gouvernement ne vise en réalité qu'un objectif de rendement budgétaire. On a beau jeu de justifier ces mesures par le soutien massif des Français à la cause environnementale, mais on ne leur explique pas que la transition a un coût, qu'il est élevé, et que ce sont eux qui la paient sur leur facture d'électricité et à la pompe. En matière de fiscalité énergétique, il est temps d'entendre nos appels à la compensation et à la modération, sans quoi vous casserez la croissance en cassant le moral des Français. Pour réduire la consommation d'énergies carbonées, il y a pour nous deux priorités priorités : le bâtiment et les transports. Dans le bâtiment, les aides à la rénovation énergétique ne sont pas à la hauteur des ambitions ; ... C'est vrai ! ... elles manquent surtout de lisibilité et de stabilité. Nous attendons en particulier depuis maintenant deux ans que l'engagement présidentiel de transformation du crédit d'impôt en prime, censée aider les plus modestes, soit tenu. Pour 2019, c'est raté, mais pouvez-vous au moins vous engager sur 2020 ? Nous pensons aussi qu'il faut mettre le paquet sur le verdissement du gaz, en favorisant la méthanisation et l'injection de biogaz dans les réseaux, ainsi que sur le soutien public aux énergies renouvelables renouvelables thermiques, notamment au travers du fonds chaleur. En matière de transports, enfin, il faut là aussi miser sur un bouquet de solutions : l'électricité pour les usages urbains, mais aussi l'hybridation, les biocarburants, le bioGNV et, plus tard, l'hydrogène renouvelable pour les transports longue distance. Il faut conclure. J'en J'en termine d'un mot sur un enjeu qui englobe tout : celui de la solidarité, non seulement envers les plus modestes de nos concitoyens, mais aussi entre les territoires. Il n'y aura

Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les sénatrices et les sénateurs, je dois d'abord vous dire que je suis très heureux d'intervenir dans ce débat. La petite histoire retiendra que ma première intervention à la tribune du Parlement en tant que membre du Gouvernement se sera faite au Sénat. J'en suis très heureux, car, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mes précédentes fonctions, je suis très attaché au bicamérisme, qui m'apparaît très utile à notre démocratie. J'en profite d'ailleurs pour saluer votre président, Gérard Larcher, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant quatorze mois en tant que président de l'Assemblée nationale. Concrètement, je souhaite travailler avec tous les parlementaires, sénateurs et députés de tous bords, qui veulent participer à la transformation écologique de notre pays. Monsieur le sénateur Gremillet, je vous remercie d'avoir fait inscrire ce débat à l'ordre du jour. Je dois dire qu'il tombe à point nommé dans notre calendrier, puisque nous allons bientôt présenter la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sera la traduction concrète de la loi de 2015 sur la transition énergétique. J'ai bien entendu votre souhait qu'il y ait une loi de programmation.

les élections présidentielle et législatives que nous nous inscririons dans ce cadre. Nous serons amenés, bien sûr, à la modifier légèrement en ce qui concerne la date, puisque mon prédécesseur et le Gouvernement ont fait oeuvre de vérité sur l'incapacité à réaliser l'objectif en 2025. En revanche, nous gardons le reste du cadre de la loi de 2015. Vous le savez, notre politique énergétique doit traduire en actes,

rétroplanning à partir de 2050 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, plus on se rapproche, plus on est dans un futur proche, plus il faut être précis. Vous n'êtes pas sans savoir que notre premier objectif,

sur l'ensemble des consommations énergétiques à l'horizon 2050. C'est évidemment un effort important, mais c'est aussi pour rappeler que l'énergie la moins polluante, celle qui n'émet pas de gaz à effet de serre, l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas.

contre les augmentations et les variations de prix. On peut critiquer, et j'y reviendrai, la fiscalité écologique, la fiscalité carbone, mais force est de constater que même si on ne faisait rien, on subirait

avec mon collègue Julien Denormandie, secrétaire d'État à la cohésion des territoires, la campagne « Faire », pour « faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique ». C'est l'outil que nous nous sommes donné pour sensibiliser les Français à l'utilité pour eux de faire des travaux de rénovation énergétique. Nous avons un objectif, vous le savez, de 500 000 logements rénovés par an. Sur la question des véhicules, nous avons aussi la volonté, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française, de réduire la consommation des véhicules, puisque, aujourd'hui, le transport routier- véhicules particuliers, camions, bus, cars -est l'une des premières sources d'émission de gaz à effet de serre. Ce n'est pas la première ! Il se trouve que nous sommes à quelques jours du Salon de l'automobile de Paris, et le Président de la République réunissait hier soir des grands dirigeants de l'industrie automobile française, européenne et même mondiale. Je participais à cette rencontre et nous avons discuté concrètement

Nous n'allons pas non plus promettre aux Français qu'il va y avoir un basculement massif vers la voiture électrique dans les cinq ans qui viennent. Ce serait quelque chose de totalement irréaliste. à l'échelle de 2050, c'est bien notre objectif d'avoir des transports qui soient totalement décarbonés. D'ici là, il faut diversifier les solutions, et je crois que nous sommes d'accord sur ce point. Cela passe à la fois par l'électrique, l'hybride, l'hybride électrique et même le gaz naturel, notamment pour les bus- c'est déjà le cas

je l'expérimente très régulièrement dans le département dont je suis issu ; en Isère, je suis régulièrement interpellé par des citoyens rassemblés en association. Alors que la très grande majorité des Français voient d'un oeil extrêmement favorable l'essor de ces énergies vertes, les élus, les collectivités qui portent ou soutiennent de tels projets se retrouvent face au syndrome au syndrome « partout, mais pas dans mon jardin ». Je souhaite plus particulièrement évoquer le sujet de la méthanisation, lequel est extrêmement prometteur, notamment pour le monde agricole. Les conclusions du groupe de travail « méthanisation », mené par Sébastien Lecornu, ont très clairement souligné tous les enjeux du développement de cette filière, pour donner aux agriculteurs les moyens de compléter leurs revenus, tout en réglant les problèmes de mise aux normes de leurs bâtiments d'élevage, et injecter une part de gaz propre, décarboné, dans le mix énergétique du pays. Des actions importantes avaient alors été annoncées. J'en rappelle quelques-unes : la mise en place d'un complément de rémunération pour les petites installations ; la facilitation de l'accès au crédit pour la méthanisation agricole ; l'utilisation des biogaz par les engins agricoles ; ou encore la mise en place d'un soutien financier pour les méthaniseurs, qui alimentent les bus

et les propositions législatives européennes en préparation viendront encore réduire la marge de manoeuvre des États. Ces derniers devront abandonner une partie de leurs prérogatives au moment même où le pilotage national semble le plus opportun. En effet, alors que le renouveau de notre mix énergétique et le déploiement des énergies renouvelables sont des priorités aujourd'hui incontestables, le mouvement de déstructuration du secteur énergétique français poursuit, sous l'impulsion européenne, certes, mais aussi par un entêtement à ne pas voir que la concurrence libre et non faussée ne peut être appliquée en matière énergétique. Nous l'avons maintes fois répété : l'énergie est non pas une marchandise, mais un bien commun de l'humanité. La privatisation de Total, le bradage de l'entreprise stratégique Alstom Énergie à General Electric, la séparation de GDF et d'EDF, le découpage d'EDF en plusieurs entités et la volonté de privatisation de l'hydroélectricité ont fragilisé le secteur énergétique français et ne permettent pas un développement cohérent des énergies renouvelables, ou ENR. Les ENR ne peuvent continuer à apparaître comme des niches profitables à des acteurs privés aidés par des subventions et par des garanties de prix de rachat payées surtout par les ménages. Cela étant, une maîtrise publique est nécessaire pour assurer la cohérence de leur développement et leur acceptation sociale, car la transition énergétique ne se fera qu'avec les citoyens. d'investir massivement dans la recherche, pour trouver des solutions aux questions de consommation, de transport et de stockage, car l'énergie de demain signera- nous l'espérons -la fin des combustibles fossiles. Dès lors, monsieur le ministre d'État, quels moyens seront mis en place afin de permettre un développement des ENR qui assure non seulement de véritables filières industrielles, pourvoyeuses d'emplois durables, des garanties collectives de haut niveau, mais aussi un prix de l'énergie accessible à toutes et tous ? La parole

ont déjà le sentiment d'être pénalisées et de supporter, plus que d'autres, le coût de la transition énergétique, d'autant que les dispositifs actuels de compensation ne sont pas à la hauteur face à la hausse de la fiscalité et du prix de l'énergie. chèque énergie est insuffisant, et la prime à la conversion pour les véhicules thermiques ne concerne qu'un très faible nombre de véhicules. Que prévoyez-vous pour que la transition énergétique soit socialement

doit être regardé comme un carburant du futur et comme un moyen efficace de stockage de l'énergie, en complément à l'intermittence des énergies renouvelables. Le « » permettra ainsi de convertir l'électricité produite et d'injecter directement l'hydrogène dans le réseau de gaz. Nous en sommes convaincus l'hydrogène vert contribuera à l'indépendance énergétique de notre pays. Une étude publiée en avril dernier estime qu'il sera en mesure de répondre à un cinquième de la demande d'énergie finale

comme le « couteau suisse de la transition énergétique ». Des initiatives jusque-là diffuses ont vu le jour et connaissent une accélération grâce à la baisse des coûts des électrolyseurs et à l'arrivée à maturité des technologies. La France doit saisir cette chance l'ont fait l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis ; elle dispose de compétences solides et d'entreprises prêtes à relever le défi. Il a fallu attendre le plan de déploiement présenté le 1 juin dernier par le Gouvernement pour qu'une véritable stratégie soit enfin élaborée. Il était temps Mais cette stratégie reste en deçà de nos attentes sur plusieurs points : faiblesse des moyens dédiés- seulement 100 millions d'euros ; manque d'ambition de l'objectif de 100 stations de distribution en 2023- l'Allemagne en prévoit 400 à la même échéance. Tout cela n'est pas très incitatif pour les constructeurs automobiles français ... Aussi, monsieur le ministre d'État, pourriez-vous nous indiquer quelle place occupera l'hydrogène dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie et quels financements seront affectés à son développement à moyen et long termes ? Il ne peut y avoir de stratégie sans visibilité !

cette taxation pèsera aussi sur les résultats des entreprises, notamment celles du bâtiment et des travaux publics. Or la pollution qu'émettent les voitures des Français ne représente pas grand-chose, si on la compare au trafic des marchandises et du transport aérien. Ainsi, le plus gros porte-conteneurs

! Pourtant, les transports maritime et aérien ne sont pas inclus dans l'accord de Paris sur le climat, et personne ne semble se soucier de ces transports extrêmement polluants.

Des entreprises privées ont évalué le potentiel de tels projets en France, et une récente étude a démontré la faisabilité de la création d'un parc de cinq lagons marémoteurs sur les côtes picardes, dans les Hauts-de-France, et sur la côte ouest de la Normandie. seules zones françaises de fort marnage dans des eaux peu profondes. La capacité potentielle d'un tel projet, évaluée à 15 gigawatts zéro carbone, permettrait de couvrir près de 5 % des besoins électriques de la France. En outre, ce projet

développement d'habitats pour les oiseaux et les animaux marins, des récifs artificiels ou des mares d'estran. Enfin, les digues qui ferment ces lagons pourraient fonctionner comme une barrière contre les aléas climatiques- tempêtes, grandes marées, etc. Elles protègeraient les écosystèmes côtiers, qui sont de plus en plus exposés au risque d'inondation et à l'érosion

Merci, monsieur le ministre d'État, pour cette réponse que je considère comme positive. Vous ne fermez aucune porte, ce qui, je crois, est à l'honneur des responsabilités que vous exercez. Je retiens votre suggestion

Monsieur le ministre d'État, l'énergie est aujourd'hui au coeur de problématiques corrélées à des enjeux majeurs, tels que la préservation de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Les questions énergétiques sont intimement liées aux mutations de nos économies et aux questions de fiscalité environnementale et énergétique. Aujourd'hui, le Gouvernement s'inscrit pleinement dans la lignée du quinquennat Hollande : une politique écologique et environnementale présentée comme ambitieuse, mais qui se résume, concrètement et trop souvent, aux prélèvements, à l'impôt, à une fiscalité de rendement. Aussi est-il urgent de reconsidérer l'équation pour proposer un énergétique consistant, maintenant qu'il y a une prise de conscience environnementale, à mettre en place en France une politique ambitieuse de préservation des ressources fossiles, de développement des énergies renouvelables et de réorientation de la trajectoire nucléaire. Pour cela, l'État doit non pas faire seul, parfois mal, mais s'associer avec tous les acteurs.

Pourquoi n'entendez-vous pas la demande que formulent les élus dans les territoires et au Parlement, appelant à une transformation de méthode dans la définition de la politique énergétique ? Quand ferez-vous le pari d'une économie décarbonée au service d'une croissance durable ? Et quels outils comptez-vous mettre en place pour relever ce défi ?

tout le monde pense qu'il faut développer les transports en commun pour permettre le basculement d'une mobilité individuelle automobile fortement émettrice de gaz à effet de serre vers une mobilité durable. Or il y faut des investissements massifs- songez au Grand Paris,

Mme Martine Filleul. Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, l'Observatoire climat-énergie a récemment publié les chiffres permettant de comparer les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone adoptés dans le cadre de l'accord de Paris

non seulement que nous ne remplissons pas nos objectifs, mais que nous en sommes loin. Ainsi, la consommation nationale d'énergie a dépassé de 4,2 points les objectifs pour

Parmi les nombreuses raisons de ces mauvais résultats figure l'absence de cohérence des politiques publiques, liée à un pilotage national insuffisant, peu efficace et peu lisible. Le Conseil national de la transition écologique a été conçu comme une instance de discussion, notamment entre l'État et les collectivités territoriales, destinée à piloter la concertation sur la transition énergétique. quand il est consulté, il peine à assurer correctement ses missions, faute de moyens humains et financiers suffisants. aucune procédure n'est prévue à ce jour pour organiser la mise en cohérence des objectifs définis à l'échelle nationale et des différents schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, territoires, ni pour réduire les effets de concurrence entre les régions inégalement dotées et mieux répartir les énergies sur les territoires.

M. Claude Kern. Monsieur le ministre d'État, dans un souci d'optimisation de la valorisation des déchets ménagers, le choix du mode de traitement de ceux-ci doit viser à tirer le meilleur parti du gisement existant. Dans ce contexte, et dans la mesure où ses impacts environnementaux et sanitaires sont aujourd'hui maîtrisés, une incinération performante reste un outil de gestion des déchets pertinent permettant de répondre à un objectif d'élimination, en y associant une valorisation énergétique. La démarche actuelle pousse d'ailleurs à valoriser au maximum l'énergie produite, en particulier sous forme de chaleur. Mais cela ne va pas sans raccordements aux réseaux de chaleur qui, paradoxalement, représentent encore une faible réalité au regard du potentiel de développement. Même s'ils sont en plein essor, la difficulté réside dans le fait qu'ils restent des outils capitalistiques : l'extension des réseaux nécessite une forte mobilisation financière, et l'amortissement se fait sur le long terme. Être performant passe par l'innovation, et les aides publiques restent en la matière un corollaire essentiel. malgré l'ambition affichée des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte- multiplier par cinq les énergies renouvelables et de récupération mobilisées par les réseaux de chaleur -, la France reste très en retard dans ce domaine.

encore faut-il, du point de vue opérationnel, que la visibilité soit au rendez-vous des investisseurs, publics ou privés. Pour les collectivités territoriales comme pour les industriels, il est donc urgent de créer un contexte de visibilité et de constance, couvrant l'ensemble des encadrements réglementaires et fiscaux.

d'État, pouvez-vous nous éclairer sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour pérenniser et favoriser le développement de ces sites d'incinération de nouvelle génération et ainsi encourager la valorisation des déchets ménagers sous forme de chaleur ?

pour les dix années à venir, le développement des réseaux de chaleur, le raccordement d'un plus grand nombre de logements et de bureaux aux réseaux seront une priorité. Il y aura une augmentation pluriannuelle

Je pense notamment à la récurrence des inondations qui ont lourdement endommagé nos communes- je l'ai vu dans mon département, la Mayenne, en juin dernier. De l'autre, on assiste à une mobilisation grandissante de la société civile et des associations, qui manifestent, alertent et attendent une traduction politique concrète de cette prise de conscience globale. De nombreux espoirs sont nés à la suite de la COP21 et de la signature de l'accord de Paris, aussi bien pour la lutte contre le réchauffement climatique que pour le nouveau modèle de croissance. Paris a toutefois une limite : malgré l'amorce d'une réflexion sur la transition énergétique, aucune des parties prenantes n'a souhaité que cette problématique soit abordée dans l'accord. On a ainsi encouragé les États à réduire leur consommation énergétique et à décarboner leur production d'énergie, sans impulser un nouveau modèle énergétique clair. De plus, derrière le problème du réchauffement climatique, d'autres questions fondamentales se posent, qui ne sont que rapidement effleurées dans le cadre des grandes négociations internationales : la pression exercée sur les ressources naturelles et la pression démographique.

pas dans cinq siècles, dans trente ans ! Cela ne peut être autre chose que la guerre ; ce n'est pas un fantasme catastrophiste, mais une analyse géostratégique élémentaire qu'il va falloir penser, nous dit cet astrophysicien. Monsieur le ministre d'État, la COP24 se tiendra en Pologne dans moins de deux mois. Alors que la France joue un rôle majeur dans la mobilisation sur le climat, quelles sont les échéances de la diplomatie française en la matière et de quels outils internationaux disposons-nous aujourd'hui pour parler de ressources naturelles, de démographie, de changement climatique et de politique énergétique

nous sommes obligés de mener une politique d'adaptation au changement climatique. Nous disposons d'ailleurs d'un plan national d'adaptation au changement climatique, que nous allons déployer. C'est absolument nécessaire pour protéger les Français

Ainsi, l'ouverture à la concurrence, consacrée voilà plus de dix ans, ne semble pas avoir atteint les objectifs attendus en matière de prix, de qualité de service ou d'accélération de la transition énergétique. Je souhaite savoir si ce ressenti est corroboré par une évaluation des effets de la libération du marché de l'énergie sur ces différentes variables. Intuitivement, on peut se demander si la mise en concurrence d'une multitude d'acteurs ne participe pas du manque de cohérence dans la mise en oeuvre des politiques énergétiques. une meilleure coordination des acteurs serait souhaitable de l'amont à l'aval, de la production à la consommation, sans oublier la gestion de l'après : je pense au casse-tête que représente dans mon département, la Loire, la dépollution et la gestion du site de l'ancienne mine d'uranium de Saint-Priest-la-Prugne. De la même manière, on peut légitimement se demander comment le domaine de l'énergie peut répondre, en même temps, à la logique de la compétitivité et aux impératifs de la transition énergétique. En effet, comment demander à un opérateur soumis à la concurrence de rechercher une limitation de sa production,

dans une certaine mesure, de l'anarchie de la concurrence et de ses abus, déjà régulièrement dénoncés par le médiateur de l'énergie. Bombardé d'informations par les marchés, le consommateur devra devenir hyperactif pour pouvoir réagir de manière rationnelle, en particulier pour s'y retrouver avec le futur contrat de fourniture dynamique. Pour répondre à ces enjeux de mise en cohérence de nos politiques et d'adaptation aux impératifs de la transition énergétique, nous avons besoin d'un plus grand volontarisme politique en matière de construction européenne de l'énergie qui ne doit pas se résumer à la construction d'un marché.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, indissociable de la souveraineté française, la politique énergétique doit concilier l'indépendance en termes d'approvisionnement, la maîtrise du coût de l'énergie et le respect de l'environnement. énergétique pour la croissance verte, la programmation pluriannuelle de l'énergie doit s'adapter aux enjeux de société et aux évolutions technologiques. Elle doit introduire dans ses objectifs principaux l'amélioration de l'efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables et la garantie de l'approvisionnement. Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre d'État, la diversification des sources d'énergie est un enjeu majeur. Or un bon mix énergétique doit garantir l'équilibre entre chacune des sources d'énergie qui présentent des qualités propres.

a bénéficié de lourds investissements, près de 160 millions d'euros, pour améliorer la captation de CO2. Elle est engagée, comme celle de Cordemais, dans un processus de transition énergétique, afin de remplacer le charbon par de la biomasse et du

serons obligés d'acheter à l'étranger l'énergie électrique nécessaire, notamment à l'Allemagne qui- paradoxe -a rouvert ses centrales à charbon.

Il faut être honnête : comme le charbon a une mauvaise image à l'échelle internationale et nationale, tout le monde trouve la décision prise assez logique. Sur les territoires concernés, c'est évidemment plus problématique, ce qui est normal : il y a des réalités humaines derrière les questions d'énergie, particulièrement quand on décide de fermer une centrale à charbon. Tout le monde parle de Fessenheim pour le nucléaire, mais on écrit beaucoup moins d'articles sur les centrales à charbon. Nous assumons ce choix, parce que, si nous voulons dire à nos voisins allemands,

La France est le leader de la production européenne de bioéthanol, avec une production de près de 12 millions d'hectolitres par an. Cette énergie renouvelable permet de réduire de 60 % en moyenne les émissions de CO2, mais elle est fortement concurrencée par des importations croissantes de biocarburants issus d'huile de palme, qui lui ont déjà pris plus de 15 % du marché en moins de trois ans. Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Pour l'instant, je constate que la modification de dénomination de la TGAP en « taxe incitative à l'incorporation de biocarburants » ne change pas grand-chose au dispositif. Le Gouvernement propose une augmentation minime du taux d'incorporation de biocarburants dans l'essence la TGAP : 0,2 % en 2019 et 0,1 % en 2020, pour un niveau total de 7,8 %, contre 7,5 % aujourd'hui, ce qui n'est pas à la hauteur de l'effort de décarbonation prévu dans les transports. La trajectoire incitative de 2017 sera dépassée de 10 % et ne respectera pas la stratégie nationale bas-carbone. Avec cette proposition, on sous-utilise le potentiel de bioéthanol pour décarboner les transports, en limitant l'utilisation de bioéthanol de résidus issus des productions sucrières et amidonnières. Or ce bioéthanol n'entre pas en concurrence alimentaire. Par ailleurs, la réglementation européenne confirme que ce produit n'est pas soumis au plafonnement européen de 7 % applicable aux biocarburants de première génération. Monsieur le ministre d'État, il n'y a donc pas de frein à augmenter plus rapidement l'objectif d'incorporation d'énergies renouvelables dans l'essence.

Nous avons en effet, en France, une filière, qui est aidée et soutenue. Nous comptons bien, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, fixer un certain niveau

au coût de cette filière qui, je le répète, s'est développée en France grâce à un certain nombre de subventions. Si cela pouvait être compréhensible pour amorcer

Monsieur le ministre d'État, depuis de nombreuses années, les différents gouvernements ont mis en avant la transition énergétique, en particulier le développement des énergies renouvelables. Les territoires essaient, malgré les difficultés, de jouer le jeu.

d'abord, il faut constater que les énergies renouvelables se développent plus vite que le réseau électrique ; ainsi, la possibilité de branchement n'est pas toujours possible. Ensuite, les gestionnaires de réseau ont des procédures de création d'ouvrages très lourdes, et donc très chronophages. Ces délais pénalisent le développement des énergies renouvelables dans la mesure où il n'est pas possible d'obtenir un raccordement dans un délai raisonnable et compatible avec la validité d'une autorisation de construire. conséquent simplifier, afin que l'ensemble gagne en agilité et en performance. En outre, le coût du branchement exorbitant et injustifié constitue une taxe démesurée. Enfin, une autre anomalie existe avec la CRE,

le ministre d'État, sur la position rigide de l'armée de l'air, qui s'oppose aux extensions, même dans les parcs existants, et ce malgré ses engagements. Or la zone SETBA, les secteurs d'entraînement à très basse altitude, touche la moitié de l'Ardèche, l'intégralité de la Haute-Loire, ainsi que le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Loire, interdisant ainsi à cet immense territoire de participer au développement des énergies renouvelables. L'exploitation des ressources naturelles représente le principal vecteur de développement économique des territoires ruraux. Ces derniers participent ainsi pleinement à la transition énergétique. La mise en place d'un parc éolien est déjà très difficile en raison souvent d'une minorité d'opposants extrémistes, mais, si l'État maintient son lot d'obstacles, elle devient franchement impossible.

M. le ministre d'État. Monsieur le sénateur Genest, vous avez tout à fait raison de souligner l'opportunité que représentent les énergies renouvelables pour notre territoire, notamment nos campagnes.

de l'éolien, vous le savez comme moi- vous êtes un homme d'expérience -, nombreux sont ceux qui se sont ingéniés à en inventer de nouveaux dans différentes assemblées, celle à laquelle j'ai appartenu pendant onze ans comme celle dans laquelle je m'exprime aujourd'hui.

En 2015, la Commission européenne a mis la France en demeure, considérant que l'attribution à EDF et le maintien à son bénéfice de l'essentiel des concessions hydroélectriques constituaient des mesures contraires à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, La France va par conséquent ouvrir à la concurrence la concession de 150 barrages hydrauliques, soit 35 % du parc national. Or nous avons l'un des seuls systèmes fonctionnant sous le régime de concession. Dans les autres pays européens, le marché hydroélectrique fonctionne le régime des autorisations, n'entraînant donc pas d'ouverture à la concurrence, d'où une absence de réciprocité. L'hydroélectricité, qui est, par définition, non délocalisable, joue un rôle essentiel dans l'équilibre du réseau électrique, répond à l'intérêt général au travers d'une contribution économique allant bien au-delà de l'aspect énergétique et, enfin, assure la protection contre les crues et la gestion de celles-ci. Alors que l'État- nous l'avons constaté en Isère -n'a pas pris ses responsabilités face au démantèlement de la branche « Hydro » de General Electric à Grenoble, filière technologique de pointe, il est primordial que notre filière hydroélectrique soit défendue, alors qu'elle nous offre une indépendance et une puissance très fortes. L'arrivée de nouveaux acteurs nous soumet à de multiples questionnements sur l'entretien de ces infrastructures, l'exigence de sécurité et les tarifs pour les consommateurs. Mais surtout, monsieur le ministre d'État, alors que la gestion actuelle concilie production énergétique et aménagement du territoire, comment sera désormais assurée la gestion des vallées, qui comportent souvent de multiples ouvrages successifs, si ces derniers ne sont pas attribués à la même entreprise ? Des risques de désorganisation et d'incohérences sont à envisager. Ainsi, qu'en sera-t-il de la sécurité des barrages et de l'approvisionnement en eau dans une situation d'éclatement des acteurs ?

EDF, le reste à la Compagnie nationale du Rhône et à la SHEM, une filiale d'Engie, autre grand groupe énergétique français.

Je ne sais pas quelle est votre position personnelle sur ce sujet, mais d'autres élus, y compris de votre département, ont tendance à plaider cela. Or le n'est pas tenable : on ne peut pas continuer avec des concessions qui sont arrivées à échéance et, donc, avec des concessionnaires qui ne savent plus s'ils peuvent investir,

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, nos débats franco-français, voire européens, finissent par nous laisser penser que le principal objectif poursuivi avec la politique énergétique est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils tiennent pour acquis le fait que nous aurons toujours assez d'énergie pour nous chauffer, nous éclairer et nous déplacer. Or satisfaire ces besoins essentiels est le véritable objet de la politique énergétique, la réduction des gaz à effet de serre étant une composante que nous devons nous imposer, mais qui a trop longtemps occulté l'essentiel. À quelles conditions pouvons-nous nous assurer que nous aurons suffisamment de sources d'énergie dans l'avenir ? D'une part, en favorisant bien sûr notre autonomie énergétique. Daniel Gremillet a montré, au début de notre discussion, que le souhait de réduire à tout prix la part du nucléaire dans la production d'électricité, alors que les énergies renouvelables ne sont pas encore tout à fait en mesure de prendre le relais, avait pour effet de dégrader cette autonomie. D'autre part, en diversifiant nos sources d'approvisionnement, ce qui permet à la fois de s'assurer de quantités suffisantes et des prix les plus bas.

naturel en énergie de l'Union européenne, qui a peu de ressources et a tendance, comme la France, à ne pas vouloir les exploiter. Nous, Français, avons tout intérêt à nous appuyer sur le plus grand nombre de partenaires possible nos voisins européens- mais les gisements britanniques et norvégiens sont limités -, le Moyen-Orient, nos amis américains et canadiens- nous avons appris ce matin le projet de Shell à Kitimat en Colombie-Britannique -et les Russes. La Russie est pour nous un partenaire stratégique en matière de fourniture de gaz. C'est le deuxième producteur mondial et le premier exportateur. Or la France et l'Europe ont intérêt à développer leur consommation de gaz

demain utilisables par le biogaz, un gaz qui ne sera pas fossile. Ces infrastructures préparent donc l'avenir. Dans l'expression « transition écologique », il me semble que le gaz peut être cette énergie de transition. Lors de notre mission, nous avons aussi constaté l'implication de nos entreprises françaises dans l'exploitation d'énergie en Russie, en particulier Total et Engie, mais aussi Air Liquide, Technip et de nombreuses autres entreprises de taille plus modeste. Engie participe au financement du projet de gazoduc Nord Stream 2 ; Total est actionnaire du premier producteur indépendant de gaz russe, Novatek, avec lequel il achève la construction d'un complexe de liquéfaction de gaz dans l'Arctique russe, sur la péninsule de Yamal. La présence en Russie de deux de nos plus grandes entreprises d'énergie est un facteur sécurisant pour notre approvisionnement, mais aussi un enjeu économique important pour notre pays. Or un obstacle se dresse quant au développement de ces activités : je veux parler des sanctions américaines prises contre la Russie à la suite de la crise ukrainienne en 2014, sanctions qui ont été aggravées en 2017 avec la question de la Syrie. Ces sanctions ont bien sûr des objectifs politiques, qui ne sont pas le sujet de notre débat d'aujourd'hui, mais elles ont des effets économiques collatéraux sur nos entreprises que nous ne pouvons pas ignorer. Depuis 2017, les États-Unis se réservent en particulier le droit de sanctionner toute entité qui participerait à un projet de, et ils mentionnent explicitement leur opposition au projet de gazoduc Nord Stream 2. Ils ont également décidé de placer Novatek sur la liste des entreprises sanctionnées. Ces sanctions américaines, prises pour des raisons de contentieux politiques, visent néanmoins de façon particulièrement forte de gros producteurs d'énergie, en particulier de gaz, comme la Russie ou l'Iran. Elles ont pour effet d'entraver l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe, au moment même où les États-Unis cherchent précisément à commercialiser leur gaz naturel issu du gaz de schiste en l'exportant par le biais des méthaniers sous forme liquéfiée. Or, pour le moment, le gaz américain est plus cher que le gaz russe, surtout celui qui est acheminé par gazoduc. De là à soupçonner nos alliés américains de chercher à fausser la concurrence à leur profit sur le marché de l'énergie, il y a un pas que, naturellement, je ne franchirai pas, mais que certains de nos interlocuteurs à Moscou ont sauté. Monsieur le ministre d'État, vous l'aurez compris, il ne s'agissait pas pour moi de dire que la France doit s'orienter vers le gaz russe, le reste du débat ayant montré que nous sommes attachés à un mix énergétique diversifié. Il s'agit surtout d'appeler à ne pas conduire une politique naïve en matière d'approvisionnement de notre énergie.

trente : Allocution de M. le président du Sénat sur les 60 ans de la Constitution de la V République. Examen d'une demande de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable tendant à obtenir du Sénat, en application de

Merci